Donc, la séance est reprise, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues lors du jour appelle les explications de vote et le vote sur la proposition de loi visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du Patrimoine présenté par Madame Dominique Vien rien et plusieurs de ses collègues.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 Sous le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues de cela a toujours été très attaché à l'action de la Fondation du Patrimoine, rien d'étonnant, me direz-vous, au regard de la mission principale qui lui est dévolu la protection du petit Patrimoine dans les territoires, le fait que cette fondation soit né d'une idée de notre ancien collègue Jean-Paul Hugot n'y est sans doute pas étranger, il est le 1er à avoir suggéré de créer une fondation privée chargée de mobiliser le secteur privé pour compléter l'action de l'État en matière de protection du Patrimoine car nous le savons tous l'État concentre l'essentiel de son action sur les monuments historiques, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui nous donne l'occasion de dresser le bilan de l'action de cette fondation et de réaffirmer l'rôle que nous souhaitons lui voir jouer dans les années à venir, aux côtés de l'État et des collectivités territoriales, c'est d'autant plus important que les années récentes ont été marquées par un nouvel élan en faveur du Patrimoine sa contribution à l'affectivité des territoires au développement économique, à la construction d'une identité locale et à la cohésion sociale est désormais clairement identifiés, c'est ce qui explique que sa sauvegarde et sa valorisation soient devenus en quelques années, de véritables enjeux de politique publique, d'où l'intérêt que la Fondation du Patrimoine puisse être aussi efficace que possible et que ces outils soient suffisamment adapté pour lui permettre l'action de l'État et des collectivités territoriales en matière de protection du Patrimoine avec son Label, la fondation dispose d'un levier d'action important pour protéger le Patrimoine qui n'appartient ni à l'État ni aux collectivités territoriales mais aux propriétaires privés, l'intérêt de ce Label est double d'une part, identifié le Patrimoine de proximité, constitué de tous les immeubles qui ne justifie pas une protection au titre des monuments historiques, mais qui est quand même présente un intérêt artistique, historique ou ethnologiques suffisant pour donner à nos territoires son café et rendre compte souhaitable sa conservation et d'autre part, encourager les propriétaires privés à le restaurer grâce à la déduction fiscale qui lui est associé et qui s'applique pour les travaux réalisés sur celui-ci mais la délivrance de ce Label est aujourd'hui soumise au respect d'un certain nombre de critères fixés par une instruction fiscale, celle-ci en a notamment restreint l'octroi à la sauvegarde du Patrimoine rural et donc principalement aux immeubles situés dans des communes de moins de 2000 habitants, d'où la proposition de Madame Veil, d'élargir le périmètre géographique du Label aux immeubles situés dans les communes de moins de 20000 habitants pour mieux couvrir l'ensemble du Patrimoine rural, mais aussi le Patrimoine non protégé urbains et industriels et permettre aux labels de contribuer aux enjeux de revitalisation des centres bourgs et centre-ville cette proposition rejoint une recommandation de la Cour des comptes qui a pas appelé de ses voeux une adaptation du Label, la commission de la culture, a accueilli favorablement ce nouveau seuil des communes de moins de 20000 habitants, tout en reconnaissant les faiblesses inhérentes à la fixation d'un seuil, il présente l'Avantage de couvrir l'ensemble du territoire Deauville à dominante rurale, ce qui explique qu'il a été retenu pour la dotation d'équipement aux territoires ruraux et pour la station de Solidarité rurale, il permet également aux labels de pouvoir être mobilisée au profit de plusieurs villes sélectionnées dans le cadre du plan Action coeur de ville ou dans le cadre du programme d'appui aux petites centralité que le ministère de la cohésion des territoires devrait lancer dans les prochains mois, la commission a supprimé toutes conditions géographiques pour la labellisation des immeubles non habitable, elle a également étendu le bénéfice du Label à l'ensemble des immeubles bâtis ou non-battu pour intégrer les parcs et jardins dans son Champ, le surcoût pour les finances publiques de ces évolutions devraient rester modérées, de l'ordre à 5 1 6 millions d'euros, ce qui n'aurait pas été le cas, si nous avions décidé de faire sauter toutes conditions d'implantation géographique l'augmentation massive du coût de la dépense fiscale qui en aurait résulté aurait non seulement été préjudiciable à nos finances publiques, mais elle aurait aussi pu fragiliser à terme le maintien de l'Avantage fiscal ce ne ont pas souhaitable au regard de l'incitation que constitue cet Avantage pour que les propriétaires engagent des travaux, notamment en ce qui concerne les immeubles non habitable, je veux dire les pigeonniers, lavoirs, les fours à pain, les puits etc, pour éviter que la protection du petit Patrimoine rural ne se retrouve marginalisés par l'extension du périmètre d'application du Label, nous avons adopté un amendement pour garantir que la moitié des immeubles labellisées chaque année appartiennent au Patrimoine rural, la Fondation du Patrimoine, nous a indiqué être en mesure de doubler le nombre de labels qu'elle délivre chaque année et s'est engagé à piloter la délivrance des labels afin d'assurer une meilleure répartition géographique aucun Label octroyé et garantir que la protection du petit Patrimoine rural reste assurée les autres articles de la proposition de loi vise, quant à eux à redonner du souffle à la fondation je souhaite plus particulièrement insisté sur l'article 3 qui réforme la composition du conseil d'administration de la fondation et on réduit l'effectif pour faciliter l'organisation des débats et améliorer la prise de décision, nous avons adopté un amendement du gouvernement qui rapproche cette composition de celle des fondations reconnues d'utilité publique, nous avons néanmoins tenu à garantir la présence d'un représentant des communes rurales au sein de ce conseil, car elles nous paraissent intéressés au 1er chef par la mission de la fondation en matière d'identification de conservation et de mise en valeur du Patrimoine de proximité, nous avons également jugé indispensable de maintenir la présence d'un représentant de l'association nationale de sauvegarde en son sein, au regard de l'appui qu'elles apportent à la fondation dans le territoire, charge à elle de s'entendre pour la personne la plus à même de représenter ce qui ne devrait pas être trop délicat puisqu'elles organisent régulièrement des réunions communes, un dernier mot sur l'article 5 qui instaure un mécanisme permettant à la fondation de réaffecter un beau votre projet de sauvegarde du Patrimoine, les sommes qu'elle a collectées dans le cadre de souscription populaire pour des projets aujourd'hui achevé ou devenu caduque et qui n'ont pas été utilisées le montant ne sont pas de négligeables, puisqu'il s'agit d'environ une dizaine de millions de francs, je sais bien que d'euros j'ai bien compris monsieur le Ministre. Que vous estimez que ce dispositif comporte des faiblesses juridiques du fait qu'il pourrait remettre en cause des contrats passés au demeurant, vous conviendrez que la situation qu'actuelle dans laquelle des dons qui ont bénéficié d'une défiscalisation sont immobilisés, plutôt que de servir la terre est générale est tout simplement inacceptable espère que vous parviendrez à nous présenter une solution juridiquement satisfaisante en 2ème lecture sur certains articles, quoi qu'il en soit, le texte qui résulte des travaux de notre commission devrait permettre à la fondation d'être plus efficace dans l'avenir, cette nous estimons que c'est dans ce domaine, l'action de la Fondation et la plus décisive, c'est un moyen de compenser la disparition de la réserve parlementaire en 2017 qui a privé des communes, en particulier des communes rurales des sauces, associations d'un outil qui contribuer chaque année beaucoup à la sauvegarde de ce Patrimoine de proximité et je vous remercie.

Monsieur le président, madame la présidente de la commission de la culture, l'éducation et de la communication Chère Catherine Morin-Desailly, madame l'auteur de cette proposition de loi chère Dominique, rien, monsieur le rapporteur, chers Jean-Pierre Leleux Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, le Patrimoine touche, nous l'avons souvent dit vous sur les bancs du Sénat moi ici à cette tribune ou dans d'autres occasions que le Patrimoine touche à ce que nous sommes, il est notre héritage commun notre lien à hier autant qu'à demain il est-ce que nous recevons et ce que nous laissons ce que nous allons laisser aux générations futures, ceux qui étaient là avant nous et ce qui restera bien après nous, il est une part de notre histoire, de notre mémoire et de notre identité, il est un levier de croissance et d'emploi de revitalisation et de cohésion, aussi, de développement et d'attractivité, nous avons pour responsabilité pour devoir de le valoriser, de le protéger et le ministère de la culture, il est engagé, vous le savez depuis maintenant 60 ans et cet engagement perdurera encore longtemps l'an prochain, mon ministère consacrera un milliard d'euros au Patrimoine au sens large, c'est-à-dire aux monuments historiques au musée, à l'archéologie aux archives L architecture dans cette action en faveur du Patrimoine, le ministère de la culture peut compter dans sa tâche dans sa mission sur des partenaires importants et je dirais même essentiel, je pense en 1er lieu aux collectivités territoriales, bien sûr, mais je pense aussi un certain nombre de partenaires comme bien sûr la Fondation du Patrimoine, comme j'ai pu le faire la semaine dernière en commission, permettez-moi d'avoir une pensée pour le président de la République Jacques Chirac et son ministre de la culture de l'époque, Philippe Douste-Blazy, car la fondation leur doit sa création la doit aussi à votre assemblée, monsieur le rapporteur, l'a rappelé tout à l'heure, elle la doit au Sénat, elle la doit en particulier au sénateur Jean-Paul Hugot qui, il y a 25 ans remettait. à mon prédécesseur à un de mes prédécesseurs Jacques Toubon un rapport sur les conditions de création d'une fondation du Patrimoine français, il y préconisait la création d'une structure de mobilisation des entreprises et du grand public en faveur du petit Patrimoine non protégé, 2 ans plus tard, cette structure devenait réalité et par la loi du 2 juillet 1996, la Fondation du Patrimoine a été crée, elle serait reconnue, elle sera reconnue d'utilité publique par décret, quelques mois après, depuis sous les présidences successives d'Édouard de Royere de Charles de Croisset et aujourd'hui de Guillaume Poitrinal, que je remercie pour leur engagement, la fondation a su développer son action en engageant des campagnes de souscription publique et des collègues de financement participatif en mobilisant le mécénat d'entreprise ou en délivrant son propre Label, en effet, dès sa création, l'État lui a confié la mission de délivrer un Label en faveur du Patrimoine non protégé au titre des Monuments historiques, celui-ci ouvre droit à un régime de déductions fiscales au titre de l'impôt sur le revenu, la fondation aussi contribué à l'initiative, plus récemment du Loto du Patrimoine, dont elle assure en lien avec mon ministère, tant au niveau des Drac, que la direction générale du Patrimoine total assure aussi donc le pilotage sélectionne les projets que la mission Bern, elle assure la gestion du fonds Patrimoine en péril donc abondé par les recettes issues du Loto du Patrimoine après 2 éditions, son succès ne se dément pas : je remercie mais non, la Fondation du Patrimoine, toutes les équipes qui travaillent, je remercie aussi Stéphane Bern qui est l'un des artisans de ce succès je remercie les Drac et les équipes du ministère en particulier, les agents de conservation régionale des monuments historiques et des unités départementales de l'architecture et du Patrimoine. En plus de leur activité d'accompagnement des propriétaires de contrôle scientifique et technique, elles fournissent un travail précieux pour la sélection des projets. En août, la Fondation du Patrimoine, a également joué un rôle capital dès le 16 avril dernier en faveur de Notre-Dame de Paris, elle est l'une des 3 fondation reconnue d'utilité publique qui ont aidé l'État opéré la souscription nationale, nous avons eu l'occasion d'en parler à de nombreuses reprises ici dans cet hémicycle, son intervention a été décisive et je veux là aussi l'en remercier aujourd'hui, fort de l'expérience qu'elle a acquise et de son modèle original, la Fondation du Patrimoine est devenu un acteur indispensable de la protection du Patrimoine dans un rapport de décembre dernier, la Cour des comptes en prend acte et formule une série de recommandations renforcer l'activité de la Fondation dans les régions où elle demeure faible faire attestée par un architecte des Bâtiments de France, ou à défaut par un délégué de la Fondation la conformité des travaux au projet instaurer une plus grande sélectivité des dossiers dans un contexte de baisse des ressources en veillant en revanche à maintenir un taux significatif de cofinancement de la fondation, améliorer la présentation comptable de l'utilisation des ressources de la fondation, plus globalement, la Cour des comptes recommande de réexaminer le dispositif du Label en vue de leur en plus efficients, elle estime qu'une simplification de la composition du conseil administration de la fondation irait également dans ce sens et Madame l', l'auteur, madame la sénatrice, la proposition de loi dont nous allons discuter s'inscrit complètement dans la lignée de ses recommandations, donc je tiens à vous remercier, madame la sénatrice veut vous êtes membre du Conseil, ministre de la Fondation du Patrimoine de l'avoir déposé, je tiens à saluer le vice-président le le qui en est le rapporteur, et qui a mené une nouvelle fois un remarquable travail de clarification du texte est remarquable travail de mise en synergie de toutes les énergies, sénatoriales et d'un travail constructif, une nouvelle fois avec le gouvernement, alors je pense en termes de clarification à la meilleure définition définition que vous avez proposé pour le Patrimoine concerné par le Label délivré par la Fondation. Je pense également à l'adaptation du code du Patrimoine aux besoins concrets, la fondation à la réalité du terrain et aux modifications introduites par la loi, et Jean vous en suis très reconnaissant, j'en profite, une nouvelle fois pour ces nains pour saluer le sénateur Alain Schmitt, délégué régional de la Fondation pour l'Île-de-France, le texte de loi vise à moderniser les outils et donc la gouvernance de la Fondation du Patrimoine alors son Label actuellement le code du Patrimoine dispose que la fondation peut attribuer un Label au Patrimoine non protégé et au site, les conditions de son octroi sont aujourd'hui uniquement définis par le bulletin officiel des finances publiques ainsi le Label peut être délivré pour 3 types d'immeubles, ce qui constitue le petit Patrimoine de proximité en zone urbaine ou rurale, il s'agit par exemple de pigeonniers de l'avoir de four à pain de chapelle de Moulins ou bien d'autres types de Patrimoine de proximité. Deuxièmement, ce qui sont les plus caractéristiques du Patrimoine rural, ils sont donc situés dans les communes de moins de 1000 habitants, ce sont par exemple des fermes, des granges, des maisons de villages, des petits manoirs ruraux par exemple et, troisièmement, ceux qui sont situés dans un site patrimonial remarquables ces critères, le texte de loi propose de les adapter les changer en nous adaptant 1er article article 1er, propose de modifier le code du Patrimoine afin d'expliciter le Champ d'application du Label. à nouveau, merci monsieur le rapporteur, pour votre effort de clarification de certains cet article puisque le Label pourra désormais être délivrés pour les immeubles bâtis ou non bâtis situés en zone rurale et et non protégés aussi des monuments historiques. Pour les immeubles situés dans les sites patrimoniaux remarquables pour les immeubles situés dans les sites classés otite du code de l'environnement et pour les immeubles situés dans des zones rurales, petite ville de moins de 20000 habitants ce réhaussement de seuil est une je pense une grande avancée et suppose en revanche davantage de moyens en faveur du Patrimoine, il était, je le sais, attendus dans le cadre des programmes de revitalisation des territoires, il est d'ailleurs totalement cohérent avec le programme Petites Villes de demain, vous l'avez rappelé monsieur le rapporteur, que le gouvernement par l'action de ma collègue Jacqueline Gourault, en lien avec Sébastien Lecornu et Julien Denormandie est en train de mettre en place et qui ciblent les villes de moins de 20000 habitants de cet article il résultera une extension importante du Champ d'application du Label. C'est donc davantage de notre Patrimoine qui sera valorisé et protégée, il faut s'en réjouir, d'autant plus que cela ne générera qu'une dépense fiscale raisonnables au regard de l'impact de cette mesure pour les territoires et pour l'économie en général, en effet, la fondation délivre environ 1000 à 1200 Label chaque année et la Cour des comptes estime que le montant des travaux réalisés par les particuliers représentent aujourd'hui 60 millions d'euros pour une dépense fiscale de 6,4 millions d'euros par an, l'élargissement du périmètre d'intervention de la fondation devrait permettre donc de doubler à peu près le volume des interventions de la fondation et ainsi le montant de la dépense fiscale qui lui être associé. Alors on a l'occasion d'en parler d'une façon très détaillée en commission mais le gouvernement émet une réserve notamment car nous continuons de penser que le taux minimum de participation de la Fondation nécessaires pour attribuer le Label doit être fixé par décret et non par la loi, mais on ne peut pas toujours être d'accord sur tout, chers amis sénatrices et sénateurs car nous considérons que ça lui permettrait d'évoluer selon les besoins, sans à avoir à changer la loi, ça peut être un risque, mais c'est peut-être aussi une opportunité de renforcer l'accompagnement financier de la fondation et surtout ceux qui bénéficient du Label 2ème point que le texte de loi propose de moderniser la gouvernance de la fondation alors l'objectif de l'article 3 de modifier la composition de son conseil d'administration pour le resserré, il paraîtrait souhaitable de rapprocher du droit commun des fondations reconnues d'utilité publique, comme le prévoit la proposition de loi la modification envisagée s'inscrit donc dans une modification plus globale des statuts, lesquels relèvent à la fois de dispositions législatives et réglementaires en vue d'améliorer la gouvernance de la fondation, le nombre de membres du conseil de ministres à Sion sera réduit les secousses crie à cet objectif, le gouvernement a proposé un amendement qui a été accepté par la commission et qui simplifie les différentes catégories de membres en retenant 3 catégories, des représentants des fondateurs mécènes et donateurs qui détient la majorité des sièges au sein du Conseil ministres Sion, conformément à l'esprit de la fondation. Des personnalités qualifiées, pouvant venir de différents horizons, des collectivités territoriales. Comme cela l'est d'usage, le nombre demandent pour chacune de ces catégories aura vocation à être définies par décret, et l'État renoncera à son pouvoir de nomination des personnalités qualifiées, elle sera désormais coopté par les autres membres du Conseil, à l'instar des autres fondations reconnues d'intérêt général. Et le président de la fondation aura vocation à être désigné parmi eux sur cette question de la simplification de la gouvernance, je tiens à remercier Jean-Pierre Leleux et les membres de la commission de la culture, l'éducation à la communication pour leur travail constructif. Comme vous, je pense qu'il est essentiel que les communes rurales continuent d'être représentés au sein du conseil d'illustration de la fondation et donc je crois que nous avons d'ailleurs mobilisés mobile modifiée, le conseil d'administration en conséquence avec la possibilité que des représentants d'associations d'élus puissent être monde. Sur cette question de simplification, je vous remercie également monsieur le rapporteur, pour votre avis sur l'article 4 en effet la possibilité pour les fondations reconnues d'utilité publique de de détenir des valeurs mobilières est désormais prévue par la loi, pacte qui a modifié la loi de 87 sur le développement du mécénat modifie. L'article 5 concerne la possibilité pour la fondation de réaffecter des dons devenue sans objet car les projets sont devenues caduques ou ont été déjà été intégralement financés en l'état sa rédaction présente des fragilités au regard du respect de l'intention du donateur, elle comporte de ce fait un risque fort d'inconstitutionnalité, elle permettra en effet à la fondation de modifier unilatéralement l'affectation des dons à certains projets sans disposer nécessairement du consentement explicite du donateur, et de celui des maîtres d'ouvrage concert. Et je redis avec force qu'il importe que le consentement des donateurs soit donné explicitement, soit au moment du don, soit au moment de sa réaffectation comme l'ont bien démontré nos échanges autour de la loi sur la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris notamment, nous mettrons, comme vous l'avez appelé à le faire, monsieur le rapporteur à profit le temps de la navette pour travailler avec le ministère de la justice et la Fondation du Patrimoine, et avec vous, a identifié une solution juridiquement adapter la difficulté à laquelle la fondation se trouver qu'on comprend parfaitement en matière de réaffectation de dons devenue sans objet car l'intention des donateurs est un principe et une garantie essentielle de l'action philanthropique et du mécénat, et encore une fois, il importe de la préserver, j'en finis Monsieur le Président, en disant que l'article 6 concerne la suppression de dispositions propres à la fondation qui n'ont jamais été mise en oeuvre, il s'agit de l'insaisissabilité, je l'ai dit de biens acquis par la Fondation pour les sauvegarder et du bénéfice d'une procédure d'expropriation au bénéfice de la Fondation et sur ces dispositions, le Gouvernement émet un avis favorable voilà Mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, la Fondation du Patrimoine et pour mon une ministère je le redis, un partenaire essentiel un partenaire indispensable et pleinement complémentaire de l'action que nous menons en faveur du Patrimoine pour gagner en efficacité, le ministère de la culture est en train de transformé, vous le savez et la Fondation du Patrimoine en a besoin, aussi, au niveau de sa gouvernance notamment, et c'est tout l'objet de la proposition de loi visant à moderniser ses outils et sa gouvernance, sous réserve de quelques différents points dont je viens de vous faire part, mais comme vous l'avez pu le constater : ils sont pour certains essentiel mais réduit dans leur nom, le gouvernement est donc favorable à son adoption. Merci monsieur le ministre, donc dans la suite de la discussion générale, la parole était Madame Mireille Jouve pour 5 minutes.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la singularité de nos territoires s'exprime à travers la richesse de notre Patrimoine local pour lequel nos compatriotes manifestent une préoccupation et un intérêt croissant les attentes à l'égard de la Fondation du Patrimoine, créée il y a maintenant 23 ans pour notamment intervenir hors du cadre des éléments classés ou inscrits comme monument historique demeure, les sénateurs du groupe du RDSE accueille donc favorablement les propositions qui sont formulées par l'auteur de la proposition de loi notre collègue Dominique verrière qui est par ailleurs membre du conseil d'administration de ladite fondation et par le rapporteur de notre commission Jean-Pierre Leleux, dont nous savons toutes ces touches la maîtrise qui est la sienne, des éléments liés au Patrimoine et à sa sauvegarde notre Haute assemblée porte aujourd'hui une réforme du Label Fondation du Patrimoine, qui est l'un des outils d'action majeure de celle-ci dans la distinction et la préservation des édifices privés présentant un intérêt patrimonial manifeste en élargissant le périmètre géographique de cette labellisation nous nous montrons notamment soucieux de nous doter d'un nouveau levier dans les efforts entrepris pour revitaliser nos centres-villes et centres bourgs leur dynamisme passe un effet aussi par leur qualité patrimoniale et l'image renvoyée par des édifices dégradés ou menaçant même ruine peut s'avérer désastreuses pour ces centres villes et bourgs en matière d'attractivité, le Sénat entend également prendre en compte une tendance de fond, au 1er janvier 2010 la France comptait désormais plus de 750 communes nouvelles cette dynamique Step révolution silencieuse comme l'évoque l'Association des maires de France, le Sénat veut l'intégrer dans sa réflexion afin de ne pas exclure du Champ de labellisation ces nouvelles collectivités dont la population, c'est c'est nécessairement accrue, nous sommes aussi conscients de l'influence que continue d'exercer certaines villes centre même de taille modeste sur leur territoire et les retombées pour ce dernier, qui est susceptible d'impliquer une valorisation du Patrimoine de celle-ci aussi en retenant désormais comme ça et de labélisation les communes de moins de 20000 habitants, nous nous efforçons de couvrir plus efficacement l'essentiel des territoires à dominante rurale afin que cet élargissement ne détourne pas la Fondation du Patrimoine de sa vocation de valorisation du Patrimoine rural, notre commission a tenu à préciser que la moitié des projets labellisés chaque année devrait s'y rattacher l'attention nouvelle portée aux parcs et jardins, nous à Paris, un autre tout à fait louable, les aménagements proposés en matière de gouvernance devrait également contribuer à faciliter la prise de décision par le biais de cette proposition de loi, la Fondation du Patrimoine voici statuts se rapprocher de ceux des fondations reconnues d'utilité publique dans le cas de la réforme de la gouvernance de la fondation, l'entrée au sein du collège des collectivités territoriales d'une représentation des communes rurales, participe de la même préoccupation de ne pas écarter la fondation de sa vocation de protection du Patrimoine rural, les nouvelles dispositions introduites relatives à la réaffectation des fonds finalement non attribuées sont aussi tout à fait opportune, il s'agit d'une manne d'environ 10 me 1000000 d'euros qui pourraient être réinjectées dans divers projets, mes chers collègues, nous savons combien les obstacles dans la protection et la valorisation de notre Patrimoine de proximité sont nombreux, ils sont avant toute chose, financier et la disparition de la réserve parlementaire est venu sur ce point encore pénaliser davantage l'action des communes, c'est au Sénat il y a plus de 20 ans que la Fondation du Patrimoine a trouvé son 1er souffle aujourd'hui sans remettre en cause la pertinence et la portée de son engagement actuel nous souhaitons lui redonner du souffle dans cet esprit de réforme, nous ne pouvons que nous réjouir de l'écoute attentive dans cette initiative, a pu faire l'objet de la part du gouvernement, l'action de proximité de la Fondation du Patrimoine est aujourd'hui indispensable pour nos territoires ruraux, même si elle ne revêt pas l'ambition d'un National Trust, le Sénat l'du fait donc oeuvre utile aujourd'hui en faisant évoluer ses outils et sa gouvernance aussi, mes chers collègues, le groupe du RDSE souscrit à la proposition qui nous est faite ce soir et votera le texte élaboré par la commission de la culture et de l'éducation ce vous remercie. Merci, la parole est maintenant à Monsieur André Gattolin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a quelques semaines nous atte tion ici même un projet de loi pour la restauration et la conservation de la 4 dalles Notre-Dame de Paris à l'époque et à ce moment-là, l'esprit de Victor Hugo, planète alors sur nos débats ce soir, c'est plutôt celui de Prosper Mérimée qui sera parmi nous poursuivons nos échanges sur cette proposition de loi visant à modernité moderniser, pardon, les outils et la gouvernance de la Fondation du Patrimoine présenté par notre collègue Dominique rien. Car si Prosper Mérimée fut un écrivain renommé, il fut aussi un archéologue très actif, je me tourne vers notre collègue Julien ce qui acquiesce et il fut surtout un défenseur acharné du Patrimoine français, au titre de sa fonction d'inspecteur des Monuments historiques, Prost, créée en 1830 et dont il exerça la fonction de 1800 son goût pour la préservation du Patrimoine se retrouve dans nombre de ses écrits, assis dans ses notes de voyage dans l'ouest de la France, adressée à l'époque au ministère de l'Intérieur, parce que je rappelle qu'à l'époque, le Patrimoine et une partie de la culture, relevait du ministère de l'Intérieur, un héritage sans doute de l'ancien régime et de sept 1er grand ministère de la culture, en tous les cas, sous autorité régalienne que fut la surintendant ce bâtiment du roi, hé bien, dans le cadre de ce voyage, il s'attarde sur l'abbaye de Beauport situé dans la commune de Paimpol, en Bretagne, en ces termes j'ai souvent eu l'occasion d'admirer la situation singulièrement pittoresque de nos vieilles des abbayes, et bien que varier à l'infini leur citons entre autres : rapport de beauté qu'il est impossible de ne pas croire que leurs premiers habitants ont éprouvé à leur aspect les mêmes sensations que nous éprouvons aujourd'hui à la lecture de ces lignes et en sachant que son auteur a fait ce qu'il a fait pour sauvegarder notre Patrimoine, il est aisé de comprendre pourquoi en 1978 lors de la création de la première base de données recensant le Patrimoine architectural français par la direction de l'architecture et du Patrimoine du ministère de la culture, celle-ci fut baptisé Mérimée le le nom de Mérimée aurait pu, avec également être attribuée à la Fondation du Patrimoine, qui a vu le jour en 1996, comme cela a été rappelé, sous l'impulsion du président Jacques Chirac et de son ministre de la Culture Philippe Douste-Blazy, reprenant en cela l'idée nos anciens collègues Jean-Paul Hugot mais aussi je veux saluer ici Yann Gaillard, mais n'en faisons point trop avec Mérimée et le Patrimoine, car chacun a sa propre lecture et je rappelle au passage, puisqu'on est dans un grand épisode culturel que Victor Hugo dans un poème qu'il consacra à la Champagne écrivit à propos du paysage de champagne ce paysage a été plat comme Mérimée comme quoi on peut avoir des visions culturelles et artistiques assez divergentes à la même époque, alors la Fondation du Patrimoine, et pour elle, a la chance de s'appeler tout simplement la Fondation du Patrimoine et c'est je crois une bonne chose, le but de la fondation et de mobiliser, on le sait, des fonds provenant d'entreprises et du grand public pour accompagner des particuliers, des collectivités ou encore des associations dans des projets de restauration du Patrimoine bâti non protégés, tels que des maisons typiques dans nos campagnes, nous en c'était un certain temps mais aussi d'anciennes usines emblématique, la fondation qui est sorti de son anonymat, on peut le dire surtout grâce au lancement du Loto du du Loto du Patrimoine en 2017 est désormais reconnu comme un acteur essentiel de la protection du Patrimoine pour améliorer son efficacité et pour élargir son Champ de l'addition, il fallait modifier quelque peu son fonctionnement et c'est ce que vous nous avez proposé chers Dominique verrière, nous avons étudié ce texte donc en législation en commission, dans le cas de la commission de la culture, la semaine passée et adopter un grand nombre d'amendements, sans rentrer dans le détail de toutes les dispositions de ce texte, j'estime que les mesures prises vont globalement dans le bon sens, c'est-à-dire celui d'une meilleure efficacité de la fondation, une démarche consensuelle élargi le périmètre d'action de la Fondation et modifier la composition de son conseil d'administration afin de Laurent de plus proche des réalités locales et de l'ouvrir à la présence d'une association nationale de protection de protection et de mise en valeur du Patrimoine, nous avons mis en conformité, le code du Patrimoine par rapport aux dispositions de la loi pacte du 22 mètres du le droit aux fondations de détenir des actions et des parts sociales d'entreprise, il appartient donc à présent à nos collègues députés d'enrichir ce texte, notamment pour trouver, comme le ministre l'a rappelé une solution juridiquement fiable quant aux sommes issus des dons à réaffecter et dans cette perspective, le groupe La République en marche votera donc en faveur de ce texte, je vous remercie. Heureusement que mes camarades sont pas là sinon je je prends cher. Bon, c'est le président, monsieur le ministre, chers collègues, la proposition de loi discutée ce soir peut sembler modeste dans ses intentions, néanmoins, ces travaux préparatoires et le rapport réalisé pour organiser notre débat dresse un bilan lucide et éclairé des missions et des moyens d'action de la Fondation du Patrimoine, plus de 20 ans après sa création, j'en remercie très sincèrement nos 2 collègues la sénatrice Dominique veut rien et le sénateur Jean-Pierre Leleux, dont la fréquentation éclairé des choses patrimonial, a donné une grande valeur aux observations de son rapport, il rappelle ainsi que la Fondation du Patrimoine avait été conçu sur le modèle du National Trust britannique mais qu'elle n'a jamais réussi à se développer avec l'ampleur de cette noble institution d'outre-Manche, les conditions de sa création, explique cet échec relatif, le National Trust a été fondée en 1895 et s'est déployée par acquisition de biens mobilisation de volontaires et extension progressive mais continue de ses missions premières dans un espace où il était quasiment seul, la Fondation du Patrimoine est au contraire une jeune institution qui a dû trouver sa place et prouver son utilité, à côté de structures plus ancienne et mieux établie, son développement est ainsi contraint par les champs de compétence, de nombreux organismes qui ont peu changé leurs pratiques à son contact, plus de 20 ans après, vous dressez, monsieur le rapporteur, un constat que je partage, il faut abandonner pour la Fondation du Patrimoine, le projet de constituer un National Trust à la française, nous devons au contraire repenser ses missions et son action en complémentarité avec celle exercée par les autres acteurs de la protection de la mise en valeur du Patrimoine, je partage l'idée défendue par ce rapport que la Fondation du Patrimoine doit prioritairement s'attacher, je cite, à l'identification à la préservation et la mise en valeur du Patrimoine non protégé, ainsi que le stipule l'article L 143 tiré 2 du code du Patrimoine par facilité administratives et parce que son statut lui permet de collecter plus facilement les fonds privés, la Fondation du Patrimoine s'est vu confier, nolens ou Lance démission pour des monuments classés ou inscrits de nombreux d'entre eux correspondent très peu à la catégorie du Patrimoine de proximité, qui aurait dû continuer à constituer le coeur de ses missions, sa participation aux aux activités de la mission de sauvegarde du Patrimoine confiée par le président de la République à monsieur Stéphane Bern a eu pour effet d'accroître cette dispersion et de l'éloigner encore davantage de son objet 1er, la Française des Jeux sera bientôt privatisée, il conviendra alors de s'interroger sur l'intérêt pour la Fondation du Patrimoine d'exercer cette fonction de portage financier pour le compte de la mission de sauvegarde, plus fondamentalement, la loi de 1996 avait confié à la Fondation du Patrimoine, a un rôle essentiel d'identification des biens mobiliers ou immobiliers ni classé et ni inscrit, il est urgent de dresser le bilan de son action dans son domaine et surtout d'évaluer comment elle a pu l'exercer en complémentarité avec les travaux réalisés par les collectivités et les services de l'État, le départ des services de l'inventaire vers les régions obligent à nous demander de quels outils nous disposons à l'échelle nationale pour apprécier notre connaissance de la variété du Patrimoine, dits de de proximité, de sa vulnérabilité et quelle politique il faudrait mettre en oeuvre pour sauvegarder parfois protégés par classement des éléments du Patrimoine qui sont aujourd'hui à la fois menacé et négligé. Lors de l'examen de ce texte en commission, j'ai cité l'exemple du Patrimoine agricole, il est composé de bâtiments de machines et d'outils qui témoignent d'une civilisation qui départ qui disparaît progressivement sous nos yeux et dont il est nécessaire de réfléchir maintenant urgemment à la sauvegarde ces actions thématiques doivent être organisées en associant tous les acteurs de la gestion du Patrimoine, les collectivités, les services de l'État et la Fondation du Patrimoine, bien entendu, la multi-cyclicité des intervenants auquel vient de s'ajouter récemment la mission de sauvegarde du Patrimoine peut conduire à une fragmentation de la connaissance et de la prise en charge du Patrimoine, cette proposition de loi et l'excellent rapport qui l'accompagne, doivent nous inciter à entreprendre rapidement un bilan de la cohérence de l'action de toutes ses institutions et de l'efficacité des dispositifs multiple d'inventaire et de sauvegarde, je vous remercie.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la sauvegarde du pape. Kim what bâti est versant essentiel de notre politique culturelle, mais le Patrimoine n'est pas exclusivement une affaire de l'État, il touche tous les Français, et bien au-delà de nos frontières, comme en témoigne la mobilisation mondiale autour de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui entend moderniser la gouvernance et des statuts de la Fondation du Patrimoine créée le la, par la loi du 2 juillet 1009. pour sauvegarder et valoriser le Patrimoine remarquables mais non protégée par la puissance publique au titre des Monuments historiques. Dans une démarche complémentaire, la Fondation apporte une réponse novatrice à la question de la protection et de la mise en valeur de plus de 400000 édifices qui forment le tissu conjonctif du Patrimoine, selon les mots de Jacques Rigaud. Elle mobilise l'ensemble des amateurs de Patrimoine en s'appuyant avant tout sur les forces individuelles des associative ainsi que sur un réseau d'entre-. Prise mécène, offrant à l'heure de sa création, une forme inédite de participation citoyenne à la vie de la cité ces leviers d'action sont de 3 ordres : la labellisation de travaux ouvrant droit à la déduction fiscale, les campagnes de souscription publique et le mécénat d'entreprise le texte que nous propose notre collègue Dominique verrions vise à moderniser le. Fonctionnement de la Fondation du Patrimoine à plusieurs niveaux, d'abord en étendant tout en limitant le Champ d'application du Label aux villes de moins de 20000 habitants. Pour un coût estimé à 5 millions d'euros supplémentaires par an, ce qui correspond à un doublement des labels délivrés, il s'agit ensuite d'élargir le Label notamment aux jardins remarquables et au parc aussi, il est prévu de réorganiser le conseil d'administration, enfin, afin de le rendre plus efficient, enfin un mécanisme spécifique permettra de réaffecter les dons, un autre projet en cas de non réalisation des travaux financés, nous partageons l'objectif du rapporteur, renforcer la mission première de la fondation, qui demeure la préservation du petit Patrimoine non protégé le plus caractéristique du monde rural, notre groupe soutient naturellement l'ensemble de ces évolutions, qui émane d'ailleurs des besoins exprimés par la Fondation elles-mêmes. Elle s'inscrit dans plus d'un siècle de mobilisation du gouvernement et du Parlement pour protéger et valoriser le pas. Les moines local remarquables qui fait la richesse de notre pays dès la période Malraux l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de France se mettait en lumière de pense oubliée des politiques patrimoniales, les Patrimoine vernaculaire et industriels au-delà du au lieu de l'histoire de France, tels que le château de Versailles, les invalides ou le Louvre, il existe disséminés dans les 4 coins du pays, d'innombrables traces remarquables d'une autre culture commune chapelle pigeonniers, lavoirs moulin ou maisons à colombages sont parfois les derniers témoins d'un monde disparu et de savoir- faire oublier. La France, pays où 90 millions de touristes n'est pas un îlot parisien cerné de vide, comme en témoigne le succès de la mission Patrimoine en péril menée par Stéphane Bern, notre identité nationale et fait de l'identité de l'ensemble des territoires. Le paysage en fait partie, les labyrinthes d'eau et de végétation de la Côte d'Opale, la Côte sauvage de Belle-Ile-en-Mer Bougival et ses impressionniste Monet, Pissarro, Renoir, sont autant de Pise paysage empreint d'une culture, d'une histoire et d'une identité propre, rappelant attention appelant le Patrimoine industriel que la proposition de loi proposait à l'origine d'intégrer dans le Champ de la labélisation constitue un autre versant oublié jusqu'aux années 1970 de notre richesse nationale anciennes tapisseries usine de fabrication de corser papeterie sites miniers raffinerie en disent long sur notre histoire sociale et sur les mutations récentes des modes de production, les tanneries et moulins du Pays de cocagne dont Toulouse, le berceau, raconte l'histoire du pastel qui sera le seul bleu portés dans toute l'Europe, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, sans entrer dans l'air du tout culturel, il ne s'agit pas de figer le passé, mais de lui redonner une seconde vie en l'intégrant pleinement au présent, moderniser la Fondation du Patrimoine c'est contribuent à cette évolution bénéfique pour nos territoires. C'est permettre à des milliers de passionnés qu'soient bénévoles, salariés ou donateurs de continuer à s'investir dans la sauvegarde du Patrimoine dans les meilleures conditions possibles, cette proposition de loi répond à une demande forte des communes, notamment celles qui se trouvent engagés dans des projets de redynamisation des centres-villes et des centres bourgs notre groupe il y apporte tout son soutien. Merci donc la parole est maintenant à Madame Dominique rien.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, quelle expérience, l'histoire de cette proposition de loi début d'un souhait de la Fondation du Patrimoine, de réduire le nombre de membres de son conseil d'administration pour le rendre plus efficace, étant moi-même administratrice au nom du Sénat ayant compris que ce qui avait été créé par la loi devait être modifié par la loi, j'ai proposé mes services et cela m'a donné l'occasion d'apprendre apprendra à mieux connaître la Fondation du Patrimoine, bien sûr, et me rendent compte si cela était encore utile de l'importance du haut de son rôle dans la sauvegarde de notre Patrimoine et particulièrement de notre Patrimoine rural apprendre à discuter certaines propositions qui pouvait mettre faite ou que je souhaitais moi-même introduire je pense entre autres aux débats sur le fameux seuil du nombre d'habitants des communes dans lesquelles le Label pouvait être accordée, je remercie d'ailleurs Catherine Morin-Desailly qui a su à ce sujet me mettre en garde contre le mieux parfois ennemi du bien apprendre comment on rédige une loi et c'est là, Jean-Pierre Leleux, que je souhaite saluer grâce à son expérience et son savoir-faire, il a su enrichir considérablement le texte pour mieux traduire nos volontés dans la loi apprendre enfin tout le travail parallèle nécessaires pour qu'une proposition de loi apparaissent dans notre agenda sénatoriales puisse être votée, qui plus est, et je vous en remercie avec un avis favorable du gouvernement. Tout un travail de discussion d'audition de débat que qui nous mène ici et maintenant dans notre hémicycle. Du travail et un peu d'sens aussi, c'est en tout cas ce que je me suis dit lorsque j'ai appris qu'outre le ministère de la culture, le ministère de la cohésion des territoires soutenait cette proposition de loi merci Jacqueline Gourault tout un travail, et peut-être aussi un peu chanceux encore je ne me cache pas pour que cette proposition de loi prospère du côté du Palais Bourbon, car il est important que cette proposition soit intégrée dans la loi, il est important que le seuil de 20000 habitants soit acté avec un doublement des labels pour aider toutes nos villes de province, à faire appel à la participation de l'action privée pour se rénover, il est important, après la disparition du Label Jardin remarquable que le Patrimoine non bâti puisse être reconnu et accompagner, il est important également que nous trouvions une solution pour récupérer les 10 millions d'euros bloqués sur les comptes de la Fondation du Patrimoine, alors que l'on sait que les projets pour lesquels ils ont été collectés ne se réaliseront pas, enfin, n'oublions pas l'objectif 1er de réduire le nombre de membres du conseil d'administration pour le rendre plus efficace. Cette réduction est un modèle d'équilibre entre les propositions du rapporteur et celle du gouvernement, elle entraîne la disparition des parlementaires du conseil d'administration, mais ce hara-kiri et le symbole de la doctrine que prône le Sénat depuis plusieurs années et la démonstration que les intérêts de Latran dation son supérieur à celui de conserver un siège une diminution, certes, mais pas sans avoir préservé la place des associations du Patrimoine et sans avoir intégré un représentant des maires ruraux ça valait donc le coup de se sacrifier. Pour autant, le Sénat ne se désintéresserait pas des activités de la fondation car notre rapporteur a prévu de leur demander annuellement un rapport sur leur activité, et ce malgré la version traditionnelle du Sénat pour ces rapports je sais donc que le travail n'est pas fini mais je sais pouvoir compter sur vos services, monsieur le ministre, pour m'aider à faire prospérer cette proposition de loi et je tiens une nouvelle fois en conclusion à remercier l'ensemble des cosignataires à remercier Catherine Morin-Desailly pour avoir accepté de l'inscrire au titre de la commission de la culture et pour ses conseils et a remercié Jean-Pierre Leleux, sans lequel le texte que nous votons ce soir ne serait pas, loin s'en faut aussi abouti et enfin je remercie mon groupe qui votera cette proposition de loi. de loi. La parole est maintenant à Madame Marie-Pierre Monier. Marie-Pierre Monier. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, un salut particulier à Dominique Verrier, un auteur de la proposition de loi, le Patrimoine sa protection et sa mise à valeur sont des enjeux qui dépassent les clivages partisans qui sont fédérateurs au niveau national comme dans nos territoires et l'examen en commission de ce texte là une nouvelle fois démontré la Fondation du Patrimoine est un acteur important du Patrimoine depuis sa création en 1996 aux côtés de l'État, des collectivités territoriales et des associations qui oeuvrent également sur le terrain, mais il faut d'aujourd'hui lui donner une un nouveau souffle, moderniser ses moyens d'action et rendre plus efficace, sa gouvernance et ses outils, les mesures que prévoit ce texte permettront en 1er lieu d'élargir les missions de la fondation est de doubler le nombre de labels qu'elle délivre chaque année pour en faire bénéficier à plus de territoire jusqu'aux petites villes de 20000 habitants, tout ce qui permet de faciliter les souscriptions et la restauration au profit de monuments qui n'étaient naguère pas concernés nous semble bien entendu tout à fait pertinent l'enjeu essentiel qui est ressorti lors des auditions et je salue le réel consensus politique il y a sur cette question et qu'avec cet élargissement, la fondation ne s'éloigne pas non plus de ce qui constitue sa mission première, la protection et valorisation du Patrimoine de proximité non protégés au titre des monuments historiques historique un Patrimoine souvent rurales, voire hyper-rural ce petit Patrimoine non classée, mais qui peut, pour présenter malgré tout un intérêt historique et artistique participe au caché au charme mais aussi à la vitalité de nos territoires ruraux plusieurs amendements proposés par le rapporteur proches des nôtres ou de nos préoccupations, qui visait à apporter un certain nombre de garde-fou, précise la rédaction de l'article 1er en renforçant la qualité du Label et surtout en garantissant que le Patrimoine rural ne soit pas la victime de acte tance extension du périmètre géographique et nous nous en réjouissons, il semblerait que le ministère des Comptes publics est accepté ce surcoût pour les finances publiques sur estimée à environ 5 millions et demi entre 5 et 6 millions d'euros, mais finalement sommes assez modérée au regard de l'importance de l'enjeu, nous resterons vigilants sur cette question du financement qui constituent le coeur du dispositif et permettrait de réelles de de réellement accroître le nombre de labels décernés annuellement et non de les déplacer vers d'autres priorités, ce qui risquerait d'être le cas si Bercy ne l'autorisait pas, pouvez-nous bien, en effet, Monsieur le Ministre, nous quand de confirmer de vive voix que il y a l'aval du ministère, des comptes publics sur ce sujet dans l'article 3 concernant la question de la gouvernance et de la composition du conseil d'administration, le texte de la commission permet de mieux prendre en compte la ruralité avec la présence des représentants des collectivités territoriales, il prévoit également la présence d'un représentant des associations de défense du Patrimoine ces 2 points satisfont ce que nous avions également défendu au travers de nos amendements, il nous paraît incontournable que ceux qui sont au plus près des projets et des territoires soit représenté si nous regrettons la suppression des parlementaires du conseil d'administration cette composition nous paraît davantage équilibré et permet en effet de se rapprocher des statuts types des fondations reconnues d'utilité publique. Je souhaiterais tout de même souligné une disposition restant dans le texte qui nous pose question, je crois que vous l'avez soulevé monsieur le ministre, dans le cas de la réaffectation non utilisés, ne nous paraît pas opportun de prévoir un d'Europe, une voie de recours en cas de désaccord entre les parties, si la décision finale revient à une seule partie en l'occurrence la Fondation du Patrimoine, cette rédaction laisse entier le problème du recours dont l'issue ne dépendrait que de la fondation, j'espère que ce dispositif n'aura pas à subir les fourches du Conseil constitutionnel, il est vrai que l'obligation de consentement Express d'un donateur pour réaffectation de son don n'est que partiellement prises en compte dans la rédaction issue de notre commission, mes chers collègues, vous l'aurez compris malgré ce petit bémol qui ne remet pas en cause l'ex-l'esprit du texte, nous voterons avec le groupe socialiste pour cette proposition de loi car les objectifs qu'elle poursuit 100 à soutenir pour la Fondation du Patrimoine pour nos territoires nos centres bourgs et nos villages. Merci, cher Merci, cher collègue, la parole est maintenant à monsieur Philippe Nachbar. Monsieur le président, monsieur le Ministre Mesdames, messieurs, mes chers collègues, les Liens entre la Fondation du Patrimoine et le Sénat sont anciens, on a évoqué tout à l'heure, le souvenir de Jean Paul Hugot, permettez moi parce que j'ai siégé avec lui au Sénat et ensemble, nous étions à la commission des affaires culturelles, telle était son nom à l'époque, lorsqu'il évoquait : d'une part, sa ville de Saumur, dont il était maire et quand on est maire de Saumur, on sait ce que représente le coût du Patrimoine et je l'entends encore dire je l'entends encore dire un jour, l'État aura beaucoup moins d'argent pour une suspension, c'est effectivement en 1995 96 il était visionnaire et c'est cette vision lucide et réaliste de l'avenir qui l'a amené à proposer la création de la Fondation du Patrimoine, il y a en France une tradition du mécénat, mais du mécénat pour le grand Patrimoine Versailles je parle sous le contrôle d'Alain Schmitt qui connaît beaucoup mieux que moi ce département Versailles a été sauvé par de grands mécènes américains mobilisés par un conservateur mais le mécénat ne s'étaient jamais intéressés au petit Patrimoine rural non-protégé comme on dit dans la nomenclature, lequel se trouvaient en situation de grand péril dans beaucoup de départements, à l'époque où la Fondation du Patrimoine a été lancée, il fallait un double dispositif : défiscalisation et bien sûr une fondation avec un statut juridiquement établie pour gérer l'argent ainsi collecté, la fondation a très vite, très vite trouver sa place, elle a joué un rôle essentiel pour le Patrimoine rural dont beaucoup, je le répète, d'éléments avaient disparu, lavoirs, fontaines, croix de mission j'appelle aujourd'hui la rapidité de la réaction, le succès des souscriptions, je peux en témoigner pour mon département, ont permis de réagir utilement je voudrais aussi saluer ici le dévouement et la compétence des bénévoles de cette armée de bénévoles qui animent la fondation dans les départements, je peux en témoigner pour le mien mais je tient à le dire d'ailleurs ici que dans un la région Grand-Est, le conseil régional a décidé de subventionner le petit Patrimoine les à une seule condition. Que le dossier soit prise en compte par la fondation qu'une souscription accompagne la subvention que le le le conseil régional du Grand-Est, je peux en témoigner puisque j'appartiens à la commission culture de cette assemblée, à condition que la Fondation accompagne le dossier et sont par conséquent la garantie de son sérieux et de son intérêt patrimonial. Elle sait parfaitement inséré dans le dispositif de la mission Bern je le dis au passage dans le dispositif du Loto du Patrimoine dont chacun ici a reconnu le succès et dans le dispositif, le ministre l'évoqué il y a un instant de la sauvegarde sauvegarde de Notre-Dame de Paris, les années ont passé et ont montré qu'il fallait compléter le dispositif, c'est l'intérêt de la proposition de déposé par notre collègue Dominique veut rien qui a pour but d'améliorer le fond dans le fonctionnement de la fondation et d'en élargir le périmètre, je ne peux que m'ont félicité, j'y vois 3 points positifs, d'abord, l'élargissement à 20000 habitants du Label qui permettra des villes petites et moyennes, lesquels ont souvent un Patrimoine tout à fait considérable dans leur centre-ville de bénéficier de ce dispositif, dont je ne doute pas un instant qu'il permettra de réussir de très belles opérations, il me paraît cependant essentiel et j'insiste sur ce point, de garantir que cette extension ne se fera pas au détriment du Patrimoine rural car beaucoup reste encore à faire dans la plupart de nos départements, il est bien de sauver les centre-villes des bourgs et des piles moyenne, il faut surtout que cela ne se fasse pas au détriment de la fondation a garantit que ces moyens, aussi bien en homme que financier qui permettrait de continuer son effort en faveur du Patrimoine rural non-protégé, je tiens à le dire ici avec force dans cette assemblée où nous avons le sens de l'équilibre des territoires 2ème intérêt l'extension du Champ d'application du Label au Parc des jardins, il avait été envisagé un temps de d'y inclure le Patrimoine industriel, il est semble-t-il maintenant indiqué déjà entre guillemets concernés par les textes, j'y attache une certaine importance, peut-être parce que je suis élu lorrain mais je trouve que nous avons dans notre pays, trop tardé à prendre en compte le grand Patrimoine industriel minier, sidérurgique textile beaucoup d'éléments magnifiques ont disparu corps et biens pour un succès comme Noisiel combien de bâtiments, dont il ne reste aujourd'hui plus rien si ce n'est quelques poutrelles ou quelques pans de murs, alors que dans les pays voisins, je pense à l'Allemagne, on a obtenu de de magnifiques réalisations en matière de Patrimoine minier et sidérurgique qui de plus grande un véritable tourisme et, par conséquent, outre l'aspect patrimonial ont un véritable, une véritable attractivité économique donc j'insiste également sur ce point, il faudra qu'on ait une politique sans doute plus actives en matière de Patrimoine industriel et puis enfin, il y a ce point un peu controversée, qui est le le déblocage de l'argent des souscriptions qui n'est pas utilisé alors que les besoins sont immenses, il est vrai que sur le plan juridique, il est un peu difficile d'imaginer réorienter des souscriptions donné pour un objet particulier je crois néanmoins qu'il est essentiel de tenter de trouver une solution à ce problème, c'est donc un excellent texte qui va dans le sens de ce qu'il faut faire pour défendre et sauver le Patrimoine sous toutes ses formes, et d'abord le Patrimoine rural non-protégé, c'est pourquoi le groupe des Républicains votera ce texte. Merci cher. Collègues Dieu donc après ces explications de vote, je mets aux voix dans le texte de la commission, la proposition de loi visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du Patrimoine, qui est pour. Qui est contre l'abstention. Donc va, proposition de loi visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du Patrimoine est adopté à l'unanimité. l'ordre du jour appelle maintenant la discussion de la proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l'art, présentée par Madame Catherine Morin-Desailly et plusieurs de ses collègues dans la discussion générale, la parole est à Madame Catherine Morin-Desailly, auteur de la proposition de loi. d'accord. En quelques instants. Monsieur le ministre reste mais Madame Madame le ministre de la justice est arrivé voilà. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. bien je je reprends, j'avais été un petit peu vite dans la transition, hein, donc, madame la ministre, madame la présidente, madame la rapporteure donc ben discussion générale de ce nouveau texte, la parole est à Madame Catherine Morin-Desailly, auteur de la proposition de loi un peu rapide. Monsieur le président, madame la garde des Sceaux. C'est le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mes très chers collègues. L'Angleterre a bâti longue pour son propre usage, la France a bâti Paris pour le monde entier, écrivait le philosophe, essayiste américain Ralph Waldo Emerson dans son journal intime, comment expliquer que la France si longtemps la patrie de la création artistique ne jouissent plus dans le domaine de l'art de la même attractivité qu'autrefois, jusqu'à la fin des années 50 notre pays occupé la première place sur le marché des ventes aux enchères, mais le marché d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier, il s'est considérablement internationalisée avec l'explosion de la demande asiatique et la vente en ligne, il tient une place de plus en plus importante, la France ne coûte plus désormais que la 4ème place, loin, très loin derrière les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni, qui mène désormais la danse dans les domaines les plus prisées, où les prix sont donc les plus élevés, je veux évidemment parler de l'art contemporain, de l'art moderne et de l'impressionnisme les atouts dont nous disposons, m'invite, malgré tout, à croire que ce déclin n'est pas inéluctable et que Paris pourrait tout à fait retrouvé la première place en Europe, qu'elle a occupé par le passé, n'oublions pas que la France reste la première destination touristique au monde et qu'elle compte sur tout le territoire, un Patrimoine aussi riche que varié, n'oublions pas non plus que la France demeure championne dans un certain nombre de domaines, tels que le Design, les manuscrits ou les arts premiers, n'oublions pas enfin que nous disposons d'un maillage étroit de maisons de ventes volontaires à travers tout le pays, dont la réputation n'est plus à faire, y compris auprès des clients étrangers, toujours est-il que ces inquiétudes autour de la perte de compétitivité de la France, nous avez conduit Philippe Bas et moi-même à prendre l'initiative d'organiser dès mars 2008 2018, pardonnez-moi de tables rondes conjointes aux membres de la commission des lois et de la commission de la culture consacré à l'attractivité du marché de l'art français, ces travaux nous avait permis d'identifier un certain nombre de blocage dont certains d'ordre fiscal, mais aussi plusieurs rigidités administratives susceptibles de Corse était le développement du marché de la en France, si elle n'a aucune prétention à relancer à elle seule la compétitivité de la France dans le marché de la ma proposition de loi très largement cosigné et je remercie les collègues m'ont fait confiance a été déposée en février dernier, elle s'inscrit dans la suite logique de ces travaux, elle vise à moderniser la régulation de ce marché et je veux remercier tout particulièrement Philippe Bas, mon collègue d'avoir demandé son inscription à l'Ordre du jour de la commission des lois, tout comme je remercie très chaleureusement Jacky de remédie en Net le rapporteur cette proposition fait également écho à plusieurs des conclusions madame Lagarde sots du rapport très approfondie d'Henriette, Chaumont et Édouard de Lamaze, que vous avez pris l'initiative de leur commander quelques mois après les travaux conduits par le Sénat en juillet 2018 si je me trompe, pour permettre à la France de retrouver sa place de leader en Europe, il faut que nos maisons et la capacité de proposer à la vente des objets de valeur, venus de France et des autres pays européens, ce qui suppose que nous disposions d'un système qui soit à la fois dynamique et qui inspire confiance, c'est ce qui justifie ma proposition de réforme du Conseil des ventes volontaires, il ne serait pas souhaitable, à mon sens, de dérégler totalement la profession, gardons à l'esprit que, contrairement à d'autres pays comme le Royaume-Uni, le secteur des ventes volontaires ne se limite pas à Paris même si c'est généralement dans la capitale que sont généralement vendus les Oeuvres de plus grande valeur, il ne faudrait pas que nous perdions ce maillage territorial si précieux, le maintien d'une instance de régulation et donc indispensable pour 3 motifs : premièrement éviter que la concentration du secteur déjà forte ne s'accroissent encore davantage, deuxièmement garantir le maintien sur l'ensemble du territoire de maisons de vente utile au tissu économique, social et culturel local, troisièmement veiller au bon fonctionnement de ce marché particulièrement exposés au risque de blanchiment et de trafic illicite pour autant je crois que le fonctionnement du Conseil des ventes volontaires n'est plus adaptée aux réalités du marché de l'art, il doit donc être modernisée, Doumé différentes propositions, tout d'abord, rebaptisé le Conseil des ventes volontaires en conseil des maisons de vente pour en faciliter l'identification. Ensuite réviser la composition du Conseil pour attribuer aux représentants des professionnels, la majorité des sièges, tout en assurant la représentation du maillage territorial et des autorités de régulation, les professionnels ne se reconnaissent pas suffisamment dans la composition actuelle du Conseil des ventes volontaires et je les comprends, alors même qu'ils sont à la base de son financement via leurs cotisations d'où l'importance d'avoir une majorité de professionnels qui permettront de tisser des Liens plus étroits avec le terrain, mais c'est également d'imprimer un esprit plus entreprenarial dans le fonctionnement de cet organe, au demeurant, j'insiste sur l'importance que tous les professionnels se sentent représentés au sein de cette nouvelle instance, quelle que soit la taille des structures ou leur implantation géographique ces évolutions qui permettront au Conseil de plus représentatifs sont de nature à mon sens, d'accroître l'écoute. Et le dialogue entre madame la garde des Sceaux, les professionnels et le gouvernement ma préposition de loi prévoit également d'élargir le périmètre des missions du Conseil pour en faire un véritable outil de concertation entre le gouvernement et les professionnels des ventes volontaires. à lui, conflit, une fonction d'information et d'observation du secteur cette connaissance est un préalable indispensable pour imaginer ensuite les outils les plus adaptés pour faire face aux différentes mutations actuelles et qui sont loin d'être négligeables quand on voit l'importance prise par les vents. Aux enchères en ligne, dernier acte de ma proposition de loi, la question des sanctions disciplinaires, un sujet essentiel si l'on veut garantir la confiance dans le secteur, la directive services n'autorise pas des professionnels, à prendre des décisions individuelles à l'encontre d'autres professionnels, d'où la difficulté de confier cette mission au nouveau Conseil des maisons de vente dès lors que les représentants des professionnels détiendrait la majorité des sièges, ce qui m'a compte nuit à proposer la création d'un organe disciplinaire indépendant au sein du Conseil des maisons de vente, composée de 3 membres, un membre du Conseil d'État, un conseiller à la Cour de cassation, une personnalité ayant cessé d'exercer depuis moins de 5 ans, l'activité d'opérateur de ventes volontaires pour éviter tout conflit d'intérêt. Je suis très attaché à cette proposition, car j'estime d'une part qu'il serait contreproductif de confier cette mission juridictions de droit commun, compte tenu de leur forts encombrements dans un secteur où il est de surcroît souvent nécessaire de statuer en urgence, d'autre part que cette option permet de favoriser la médiation, ce qui paraît devoir être privilégiée dans un secteur comme celui-ci, j'espère Madame la garde des Sceaux, que l'examen de cette proposition de loi se poursuivra dans les quelques semaines à l'Assemblée nationale, tant nous sommes nombreux à partager le constat de la nécessité de légiférer en la matière et parce qu'il faut également répondre à une profession qui est depuis qui est depuis longtemps dans l'attente je ne doute pas qu'elle puisse servir de base de discussion et que nous parvenions à trouver des points de convergence au cours de la navette pour lui permettent de connaître le même destin qu'une autre proposition de loi. Sénatoriales voté ces dernières semaines à l'unanimité de lots de sang je pense bien sûr à la proposition de loi que nous et vieux qui ont quelques instants avec le ministre de la culture, instaurant un droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse, je vous remercie de votre attention. Merci, la parole est maintenant madame Jacky Deromedi, rapporteur de la commission des lois. Monsieur le président, madame la garde des Sceaux, monsieur le président de la commission des lois, madame la présidente de la commission de la culture, mes chers collègues, la commission des lois a examiné avec beaucoup d'intérêt cette proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l'art, déposée par la présidente Catherine Morin-Desailly à la suite des auditions organisées conjointement par nos 2 commissions sur la situation du marché de l'art français en mars 2018, ce texte a pour objet de réformer notre système de régulation des ventes volontaires de meubles aux enchères aux enchères publiques dans la vente d'objets d'art et de collections représentent environ la moitié comme vous le savez, ce secteur d'activité a été progressivement libéralisé depuis le début des années 2000 avec l'abolition du monopole des commissaires-priseurs, la suppression de leurs offices ministériel et le passage à un régime d'agrément, puis un simple régime de déclaration préalable des opérateurs certaines pratiques qui contribuaient à l'acte, tracts, éviter des maisons de vente étrangères mais qui était naguère, prohibées en France ont par ailleurs été autorisé, comme le prix de réserve la garantie de prix, les avances sur le prix d'adjudication, les ventes after ou encore la vente aux enchères de biens neufs dictée par la nécessité de mettre la loi française en conformité avec le droit européen, ces réformes ont également eu pour ambition de rendre son lustre d'antan au marché français dans les années 50 en effet, la France se situe au 1er rang mondial pour les ventes aux enchères de meubles, elle n'est plus qu'au 4ème rang, loin derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et désormais la Chine sur ce terrain, la libéralisation n'a pas eu les effets escomptés, même si le volume total des ventes aux enchères réalisée en France a progressé, cela n'a pas suffi à rattraper notre retard par rapport aux champions mondiaux dans le seul secteur des objets d'art et de collection, on estime que la part de marché de la France stagne autour de 6 pourcent du marché mondial, en outre, pour beaucoup d'anciens commissaires priseurs, la perte de leur monopole d'officiers ministériels sur l'activité de vente volontaire et et la soumission de cette activité au contrôle d'un organe de régulation extérieurs à la profession ont été difficiles à accepter la proposition de loi dont nous sommes aujourd'hui saisies a pour principal objet de réformer cet organe de régulation, le Conseil des ventes volontaires en modifiant sa composition Son organisation interne, ses missions et, jusqu'à sa dénomination à titre préliminaire, nous devons nous interroger : est-il pertinent de maintenir une autorité de régulation propre au secteur des ventes volontaires de meubles aux enchères qui constitue une singularité française, ce n'est pas certain. Sans doute l'activité de vente aux enchères doit-elle être soumise à une réglementation, sans doute, des contrôles sont-ils nécessaires pour éviter les risques de fraude liés au procédé des enchères, ainsi que les risques de recel et de blanchiment particulièrement élevé dans le secteur du marché de l'art néanmoins ces contrôles pourraient être du ressort de services ministériels, financée par l'impôt, comme c'est le cas d'autres activités présentant le même genre de risques j'ai toutefois plus constater au cours des auditions que j'ai conduite qu'il n'existait aucun consensus pour s'engager dans cette voie, ni parmi les professionnels, ni parmi les administrations compétentes pour beaucoup le indien, le maintien d'une autorité de régulation Haddock est non seulement indispensable pour protéger efficacement les vendeurs et des acquéreurs, mais c'est aussi le moyen de préserver l'image très positive dont jouissent les maisons de ventes françaises à l'étranger, en d'autres termes, un système de régulation plus rigoureux en ce qui garantit la sécurité des ventes et prémuni contre les fraudes peut aussi constituer un Avantage on comparatif dans un marché mondial très compétitif, la commission des lois a donc approuvé la loi la voie médiane choisie par nos collègues qui consiste à réformer en profondeur l'Autorité de régulation sans la supprimer, bien entendu, cette réforme, à elle seule ne suffira pas à rendre son dynamisme au marché français des enchères, il serait d'ailleurs présomptueux de prétendre y parvenir par la loi, le déclin du marché français à des causes multiples : outre une réglementation qui fut longtemps très restrictive, outre le poids des contraintes administratives et fiscales ce déclin, c'est s'explique aussi par des facteurs sur lesquels le législateur à moins de prise des facteurs culturels, d'abord, Paris n'est plus comme autrefois la capitale mondiale des Beaux-Arts des facteurs sociaux socio-économique, ensuite les acheteurs les plus fortunés vivent aujourd'hui à l'étranger, par ailleurs, comme le souligne le récent rapport remis à Madame la Garde des Sceaux par Madame Henriette bon et Me Édouard de Lamaze, il est indispensable de promouvoir un esprit plus entreprenarial au sein de nos maisons de vente afin qu'elle sache s'adapter mieux encore aux attentes et aux besoins des consommateurs, il n'en demeure pas moins qu'une autorité de régulation plus à l'écoute des professionnels pour les aider à réussir leur mutation. La commission des lois, donc source a donc souscrit à la proposition tendant à ce que les représentants de la profession soit désormais majoritaire au sein du collège de l'Autorité de régulation rebaptisé Conseil des maisons de vente et s'est contentée d'apporter divers ajustements omission à la composition à l'organisation et au fonctionnement du nouveau conseil, en outre, la commission des lois a complété le texte en y ajoutant plusieurs dispositions de nature à stimuler l'activité des maisons de ventes françaises, ainsi nous avons étendu aux meubles incorporels le régime légal de vente de meubles aux enchères, ce qui permettra à nos maisons de ventes de développer de nouveaux marchés, par exemple pour la mise en aux enchères de fonds de commerce, nous avons ouvert la voie à ce que les maisons de vente puisse réaliser certaines ventes aujourd'hui considéré comme judiciaire est réservé aux officiers ministériels, bien qu'il ne s'agissait pas de vente forcée, je pense par exemple à la licitation de biens de succession, nous avons créé les conditions d'une concurrence équitable entre d'un côté, les maisons de vente de l'autre côté les officier public ou ministériel habilité à réaliser des ventes volontaires, à savoir les notaires et les futurs commissaires de justice nous avons allégé le poids des procédures en réduisant le formaliste dès le formalisme des ventes de gré à gré et en autorisant le regroupement du livre de police et du répertoire des procès-verbaux, enfin, nous avons souhaité que les personnes physiques habilité à diriger des ventes volontaires retrouve le beau titre de commissaire priseur aussitôt que la profession de commissaire-priseur judiciaire aura disparu, pour être regroupées avec celles d'huissiers de justice, si cette proposition de loi ne constitue pas une révolution, je suis convaincu qu'elle redonnera un souffle aux maisons de ventes française et à mieux les armées pour faire face à la compétition internationale, toutefois, comme le soulignait le rapport Chaumont le le Hamas leur rêve, leur avenir est en grande partie entre leurs mains, je vous remercie. Merci, la parole est maintenant Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la justice. Monsieur Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure j'quitté remédie mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, depuis plusieurs mois, la question du marché des ventes volontaires a suscité beaucoup d'attention de la part des parlementaires le texte dont vous allez débattre aujourd'hui à l'initiative de Madame la Présidente Morin-Desailly que je salue particulièrement en témoigne, tout comme d'autres propositions également intéressantes qui ont été portés à l'Assemblée nationale, de son côté, le gouvernement et au 1er chef mon ministère ont également été très attentif à cette question en travaillant très étroitement avec les professionnels du secteur, je me réjouis donc de l'examen aujourd'hui de ce texte dans votre hémicycle, je m'en réjouis, parce que vous vous saisissez et madame la présidente, et Madame la rapporteure l'ont dit, vous vous saisissez d'une question importante : comment renforcer l'attractivité et la compétitivité juridique du marché de l'art français, la France dispose d'atouts tous indéniable sur le marché de l'art, la richesse formidable et inégalée de son Patrimoine, les compétences et la formation des professionnels, ainsi que l'ancrage territorial des sociétés de vente volontaire en dépit de ses atouts, les professionnels comme les représentants des instances de régulation et de contrôle, déplore pourtant un certain déclin de la place de la France en cette matière, il est donc apparu nécessaire pour préserver l'attractivité économique de la profession de réfléchir à son adaptation aux importants défis auxquels elle doit faire face à ces défis sont au moins au nombre de 3 : l'internationalisation, la concentration du marché et la numérisation votre assemblée dès le mois de mars 2017 s'est saisi de cette problématique lors de plusieurs auditions qui ont été menées par vos comités, commission des lois et de la culture précisément sur l'attractivité et la compétitivité juridique du marché de l'art français, j'ai moi-même perçu l'urgence et l'inquiétude des professionnels : en raison de l'arrivée sur le marché, d'autres acteurs et d'une concurrence internationale croissante, mais aussi en raison des conséquences de la réforme des commissaires de justice, c'est dans ces contextes, comme vous l'avez rappelé madame la rapporteure, madame la présidente, que j'ai confiée Henriette bon Édouard de Lamaze, en juillet 2018, une mission sur l'avenir de la profession d'opérateurs de vente volontaire. Le texte que vous présentez aujourd'hui rejoint en partie les propositions du rapport qu'ils m'ont remis en décembre 2018 comme je veux souligner d'emblée ces propositions ont également suscité l'attention des élus du Palais-Bourbon, ainsi le député Sylvain Maillard et le groupe La République en marche, avec notamment le député Jean-Michel Miss ont déposé une proposition de loi sur ce sujet avec plusieurs échanges avec la chancellerie tout au long du printemps vous 2 propositions de loi traduisent un consensus auquel je m'associe, autour de l'indispensable réforme de la réglementation de la profession pour faire face aux défis auxquels elle est aujourd'hui confronté à l'évidence, la proposition que vous allez examiner s'inscrit dans le sillage du mouvement de libéralisation des ventes aux enchères publiques, qui a connu 2 réforme de grande ampleur, l'une en 2000 et l'autre en 2011, ces 2 grandes réformes ont façonné l'exercice de cette activité séculaire pour s'adapter à une nouvelle donne. La loi du 10 juillet 2000 que vous avez évoquée, a mis fin au monopole des commissaires-priseurs, elle a établi une distinction entre d'une part les ventes judiciaires prescrites par la loi ou par une décision de justice qui relève de la compétence des officiers publics ministériel et d'autre part, les ventes volontaires pour assurer ses ventes volontaires ont été créées, des sociétés de vente volontaire soumise à l'agrément et au contrôle disciplinaire du Conseil des ventes volontaires, la loi du 20 juillet 2011 pour sa part, a tiré les conséquences de l'adoption d'une directive européenne, celle du 12 décembre 2006 relative au service dans le marché intérieur, c'est la directive Services, cette loi à apporter des innovations importantes qui se sont traduites par un assouplissement dans le fonctionnement des structures professionnelles par une extension du Champ d'activité des opérateurs et par une diversification de leurs modes d'intervention, mais parallèlement à ces évolutions juridiques, le marché de l'art, je le disais tout à l'heure, a fortement muté sous l'influence d'une internationalisation de plus en plus grande, et d'un développement des ventes non régulée en ligne. Ces bouleversements ne sont pas sans conséquences sur la double exigence et de protection des usagers acheteurs comme vendeurs et de compétitivité du secteur ainsi que l'écrivent Henriette chaud bon Édouard de Lamaze et je les cite en termes économiques la libéralisation totale du marché, et sa dérégulation placerait les professionnels des ventes volontaires selon le phénomène de ciseau dans une situation de concurrence intenable avec d'un côté, les 6 turcs commissaire de justice et de l'autre les maisons anglo-saxonnes, les rapporteurs en ont donc conclu qu'au sein d'un marché libéralisé le maintien d'une instance de régulation propres à assurer son bon fonctionnement à vérifier sa transparence et le respect des garanties qu'il doit offrir à protéger les vendeurs et les acheteurs et à veiller aux bonnes conditions d'exercice de l'activité par ces professionnels, cet organe de régulation était indispensable. Un consensus donc se dégage aujourd'hui sur la nécessité pour le secteur des ventes volontaires de parvenir à relever 3 défis principaux accroître l'attractivité et la compétitivité des maisons françaises sur le marché mondial, préserver la sécurité et, par là même la pérennisation des ventes volontaires aux enchères publiques favorisé, enfin, l'accompagnement des professionnels et la protection des consommateurs, l'une des lignes de force du rapport ce de la masse repose sur l'idée qu'il ne faut pas voir dans la réglementation actuelle, un frein à l'activité des ventes volontaires je souscris pleinement à cette idée, qui traduit d'une certaine manière, les exigences que vous portez vous-même dans la présente proposition de loi, au contraire, cette réglementation est un gage de sécurité, de transparence, d'objectivité dans la valeur du bien et la détermination des prix elle concourt également et j'ai été très attentive au fait que vous relevez Vier ce point-là elle concourt également à la préservation du maillage territorial et c'est un point auquel je suis également pleinement attachés, ainsi d'ailleurs, qualité d'image d'excellence de la France en la matière. La présente proposition de loi poursuit donc le réforme la pardon, le mouvement de réformes engagé par les textes précédents et concilie une plus grande liberté sur le marché des ventes volontaires avec le nécessaire maintien d'une régulation gage de crédibilité et de probité dans un secteur qui impose une véritable attention et une très grande rigueur au regard des risques de fraudes qui peuvent le traverser. La libéralisation de la profession de commissaire-priseur en 2000 a conduit à la création du Conseil des ventes volontaires devenu en application de la loi du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, l'Autorité de régulation de ce secteur, le rapport toujours de Madame Michaud bon et de Me de Lamaze relève que si le Conseil des ventes volontaires et parfois critiquée, notamment quant à sa composition, il permet néanmoins d'assurer la crédibilité et la confiance dans le marché des ventes volontaires, le principe d'une régulation et donc je le redis, indispensable pour éviter que la concentration ventes concentration qui est déjà forte ne s'accroissent davantage et pour garantir le maillage territorial des maisons de vente qui constitue un atout économique, social et culturel tout à fait considérable le consensus qui se dégage aujourd'hui sur la nécessité de moderniser le Conseil des ventes volontaires étaient réelle parce que ce conseil ne correspond plus, vous l'avez dit, madame la présidente, madame la reporte la rapporteure ne correspond plus au réalités du marché, le texte que vous allez examiner vise donc à moderniser la composition du Conseil des ventes volontaires ces missions, son financement et le volet disciplinaire de la profession quant à la composition, le texte prévoit que le Conseil des maisons de vente nouvellement dénommée soit composé d'une majorité de six, professionnels, élus et de 5 personnalités qualifiées nommées respectivement par le garde des Sceaux, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du commerce, cette composition répond à à la volonté des professionnels d'une présence accrue au sein de l'organe de régulation, tout en assurant la représentation du maillage territorial, je suis favorable à ces orientations qui me semble traduire les besoins et les attentes de la profession afin toutefois de préserver l'équilibre entre le caractère professionnel du Conseil et sa fonction de régulation je vous proposerai un amendement visant à ce que le président du Conseil soient désignés par le garde des Sceaux, parmi les personnalités qualifiées et non parmi les professionnels en effet associée à une présence majoritaire de professionnels, la nomination du président parmi ces professionnels rapprocherait selon moi cette autorité de régulation d'un ordre professionnel, ce qui n'est pas l'objectif de cette réforme et ne m'apparaît pas souhaitable au regard de l'équilibre recherché afin d'assurer l'ancrage dans les territoires, je vous proposerai également au nom du gouvernement un amendement traduisant dans la loi la diversité territoriale des opérateurs de ventes volontaires parmi les professionnels, élu au sein du Conseil des maisons de vente. Votre proposition de loi conserve par ailleurs les redéfinissant les missions actuelles du Conseil des ventes que sont notamment l'identification des bonnes pratiques et l'élaboration d'un recueil d'obligations déontologiques, l'observation de l'économie des enchères, l'organisation de la formation professionnelle, mais votre proposition complète ses missions par des missions nouvelles, je les cite, information des professionnels et du public sur la réglementation applicable soutien et promotion de l'activité des ventes volontaires prévention et conciliation des différends entre professionnels, examen des réclamations dirigée contre les opérateurs. S'agissant du volet disciplinaire, la proposition de loi s'inspirant des propositions du rapport chaud bon de Lamaze institut un collège une commission d'instruction une commission des sanctions, je note que la proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par messieurs par monsieur Maillard propose quant à elle, le transfert de la discipline aux juridictions judiciaires, ce qui au regard du faible nombre de contentieux actuellement traité et peut-être une option plus simple, la navette parlementaire permettra d'avoir un débat sur cette question primordiale pour la crédibilité du secteur de vente volontaire je souhaite ici avant de terminer et rendre un hommage au travail effectué par Madame la Présidente Morin-Desailly et par Madame, la rapporteure de remédie je ne doute pas qu'un travail fructueux d'enrichissement de cette proposition sera menée dans le cadre de la navette parlementaire que j'évoquais et contribuera à renforcer l'attractivité de la profession au service de la tradition française d'excellence en matière de vente volontaire, je voudrais simplement pour conclure préciser que, au-delà des évolutions structurelles qui sont proposés dans le texte que nous allons étudier maintenant le rapport chaud bon de l'Amazone qui n'ignore pas que le marché les ventes volontaires présente un certain nombre de caractéristiques qui sont autant de fragilité propose un certain nombre de mesures pour identifier les marges possibles de progression un certain nombres de ces mesures relève de de du domaine législatif, d'autres du domaine réglementaire, pour ma part et à vos côtés, je mettrai tout en oeuvre pour que l'ensemble de ces dispositions viennent redonner souffle et assure une longue vie au maison de vente volontaire et au commissaire-priseur, je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Entre dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur André Gattolin.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est à l'initiative de notre collègue Catherine Morin-de me que nous débattons aujourd'hui de cette proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l'art plus largement que ce que son intitulé veut bien laisser deviner ce texte vise l'ensemble des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, composé d'un article unique, la PPL d'origine prévoyait la transformation du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en conseil de maisons de vente, l'objectif : donner plus de liberté aux maisons de vente créer un organe disciplinaire indépendant mais également mettre en place une instance chargée de représenter les professionnels auprès des pouvoirs publics, cette proposition, disons-le sans aiguille ambiguïté était attendue des professionnels et les donc salué par eux, mais elle est également le fruit de plusieurs rapports qui concluait à la nécessité de réformer le Conseil des ventes, je n'ai très puisque ça n'a pas été fait jusqu'à présent, le rapport de Stéphane Travert de novembre 2016 sur le marché de l'art, et bien évidemment le récent rapport Chevron Lamaze, qui vous a été remis l'an dernier, madame la garde des Sceaux, la commission des lois du Sénat tout en approuvant les grandes lignes de cette réforme proposée de l'organisation interne de cette autorité a apporté quelques modifications substantielles, notamment en recentrant l'activité du conseil sur sa mission de régulation, elle a également précisé sa composition, je crois, à ce titre que l'amendement déposé par le gouvernement sur la représentation territoriale des opérateurs de ventes volontaires parmi les professionnels, élus au sein du Conseil est un amendement de concernant le régime disciplinaire, la commission des lois également clarifier les règles applicables au fonctionnement de la commission d'instruction tout d'abord, en précisant que la commission d'instruction devait constituer un organe distincts de la juridiction disciplinaire, puis dans son organisation en précisant les règles applicables en cas d'empêchement ou de départ simultané de membre titulaire ou en cas de désaccord entre 2 membres de la commission, en résumé, mes chers collègues, ce texte attendue et saluée par les professionnels des maisons des ventes est relativement consensuel, à ce titre, le groupe La République en marche le soutiendra en attendant naturellement que nos collègues députés le débat et l'enrichisse à leur tour, il ne faut cependant pas se leurrer sur l'un de ses s'objectif qui est de l'inscrire dans une stratégie plus globale de reconquête du marché de l'art mondial réformer la régulation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Nora il faut bien se l'avouer qu'une incidence secondaire, voire minime sur la place de notre pays sur le marché de l'art, l'essentiel du marché de l'art aujourd'hui, on le sait, a lieu dans 3 pays : le Royaume-Uni, les États-Unis et la Chine, qui assure environ 90 pourcent du chiffre d'affaires global la part de la France ne représente en moyenne qu'environ 4 pour 100 de celui-ci, les principales ventes en 2019 ont lieu à New York ou à Londres et, malgré les ventes record sur l'art moderne, les maisons françaises n'en profite pas le déclin de Paris, il faut le dire, a commencé dès l'après-guerre à l'époque de était encore le principal lieu de vente dans le monde et son chiffre d'affaires était équivalent à celui de Sotheby's et de Christie's réunis le recul de la France, c'est définitivement durant les années 60 Jean Cordier qui était Compagnon de la Libération et ancien secrétaire de Jean Moulin avait assez bien résumé la situation lorsqu'il ferma sa galerie en 1964 en 10 ans Paris fait désormais partie de la périphérie par rapport à New York depuis ces 20 dernières années, la montée des places asiatiques n'est pas étrangère à l'enrichissement rapide de la région, et notamment de certains hommes d'affaires ou responsables chinois pourtant mes chers collègues, nous avons aujourd'hui une belle opportunité de mon ou de reconquérir des parts de marché mondial de l'art, grâce aux effets à venir du Brexit et des des galeries actuellement ferme à Londres tandis que de nouveaux espaces ouvre à Paris, notre point fort, c'est le marché unique, nous devons en profiter pour nous demander pourquoi le chiffre d'affaires des maisons de ventes française est si faible et comment il est possible d'augmenter le volume des ventes, faut-il simplifier le fonctionnement des maisons de vente faute simplifier l'accès à la profession de commissaires-priseurs volontaire, comme le préconise le rapport bon la de Stéphane Travert j'revient l'a très bien dit, le statut et le monopole des commissaires-priseurs a conduit une démarche de contournement du marché français, les maisons de vente étrangères qui se sont sentis exclus de notre pays par la réglementation française ont développé en réseau et des outils tellement performant que le retard pris peut parfois paraître irrattrapable mais plus encore que la réglementation, je crois que l'axe sur lequel il faudrait collectivement avancé et celui de la scène française et de la création artistique, je dis collectivement parce qu'en 1er lieu nos institutions comme nos collectionneurs doivent oser mettre en avant des artistes français si François Pinault ou Bernard Arnault sont des collectionneurs influents, ils le sont grâce à leurs achats internationaux mais à l'exception de Daniel Buren, il ne mettent pas en avant des artistes français alors acheter français en la matière ne se décrète pas, il y a donc, je crois encore beaucoup à faire, notamment en association notre ministère de la culture et nos grands acteurs économiques et financiers pour redonner tout son lustre à notre pays sur le marché de l'art, je prends merci. Merci, la parole est maintenant à Madame, Esther Benbassa.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, la France possède une culture Childish pluri-séculaires et probablement l'une des plus belles au monde, elle est un haut lieu dollars depuis la renaissance, et Paris a longtemps tenu comme mes collègues l'ont déjà dit, la première place du marché de l'art mondial depuis les années 1960 le marché de l'art français et pourtant sur le déclin avec 5 à 6 pourcent de parts de marché à l'échelle mondiale

les raisons en sont multiples et touchent au domaine artistique, fiscales, administratives. Premièrement, artistique, car la France n'arrive plus à produire suffisamment de correspondant aux attentes du marché mondial de la sa politique culturelle se détourner de l'art pictural pour embrasser à partir des années 1980 un art conceptuel qui n'a trouvé que relativement peu de débouchés sur la scène mondiale. Deuxièmement fiscale car la France n'a pas mis en place des mécanismes suffisamment incitative pour que le mécénat viennent compenser l'investissement public. à partir dans le à partir de là, de ces dernières décennies, la loi Aillagon de 2003 était pourtant venu et réformer les modalités des dons des particuliers du mécénat des entreprises et de la fiscalité des fondations, mais de toute évidence pas suffisamment pour que le secteur privé, assure le maintien d'une véritable politique culturelle de qualité là où l'État se faisait défaillant. Le Conseil des ventes volontaires posent un problème de taille dès sa création en 2011, le groupe CRCE avait alerté sur les problèmes que pouvaient causer une autorité de régulation venant libéraliser le marché de la cette mesure avait permis de faire la part belle aux grandes maisons de vente mondialement célèbres au détriment des petites maisons françaises, cette proposition de loi pour mérite de vouloir renforcer la présence des professionnels du marché de l'art au sein du CV, la situation devrait ainsi servir à faire le lien entre les artistes et les autorités de régulation à l'image du ministère de la culture, on peut s'interroger sur la jonction à vouloir faire de Paris une place prime primordial sur le manche, marché mondial de l'en effet le tissu artistique français si spécifique Laurent peut-être antagoniques Haïm vision libérale et concurrentielle surtout gagner une place de choix tant prisée sur le marché mondial ne garantit pas une prospérité économique pour des centaines d'artistes français qui n'arrivent pas aujourd'hui à joindre les 2 bouts, nos artistes doivent pouvoir vivre de leur travail et soutenu dans ce sens, pour ce faire, la France possède un potentiel hors du commun, sa capitale dispose d'un démaillage de galeries d'art les plus denses au monde et le savoir-faire de ses musées reconnu internationalement, au point que certains d'entre eux possèdent des antennes culturelles à l'étranger, à l'image du Centre le Pompidou à Shanghai ou encore du Louvre d'Abou Dhabi, accroître le rayonnement culturel de la France dans le monde est certes un objectif souhaitable mais pas suffisant ainsi devant nous valoriser nos filiales artistique permettent l'émulation saine handball nos jeunes talents par la création d'un concours national, à l'image du canal prend britannique met en place encore plus d'événements dédiés à la sur le modèle de ce que nous faisons pour le cinéma à Cannes ou faut la BD Angoulême exigeant également l'Exposition de plus d'artistes français d'art contemporain dans nos musées, pour l'heure, seule réforme de grande ampleur, permettre à la France, c'est de retrouver son influence d'antan, le présent texte contient un ensemble de dispositions intéressantes mais bien timorés qui ne se ne suffiront pas à réaliser, c'est objectif en l'état, le groupe CRCE s'abstiendra merci. Merci donc la parole est maintenant Madame Colette Mélot. monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à moderniser la régulation du marché des ventes aux enchères publiques opérée par le Conseil des ventes volontaires rebaptisé Conseil des maisons de vente, l'existence de cet établissement est une particularité française, si bien que la question de sa suppression est souvent évoquée au profit de la création d'une Direction dédié à ce secteur au sein du ministère de la culture, l'auteur du texte, la présidente Catherine Morin-Desailly, ainsi que la rapporteure notre collègue Jacques Hydro-Mehdi, dont je salue le travail, on fait le choix de préserver le Conseil des ventes volontaires tout en proposant une réforme de fond visant à moderniser l'établissement, il s'agit pour l'essentiel de renforcer son efficacité, la transparence de son fonctionnement et d'agrandir son périmètre d'action. La commission des lois a souhaité recentrer ses missions sur la régulation du secteur, en supprimant la proposition de doter le Conseil d'une fonction de représentation des opérateurs de vente volontaire auprès des pouvoirs publics publics rôle réserve Nous saluons également l'adoption d'un amendement visant à autoriser l'établissement à effectuer des contrôles sur place, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, selon les estimations du FMI, le marché noir des Oeuvres 10 Oeuvres d'art représenteraient en 2019 un volume de 6 milliards d'euros, soit 10 pourcent du marché de l'art, ces pratiques sont renforcés par l'opacité du marché et l'anonymat des acheteurs qui devrait être levée pour les transactions supérieures à 10000 euros en application dès janvier prochain de la 5ème directive européenne antiblanchiment. La création d'un organe disciplinaire distincte du Conseil contribuera également à renforcer l'efficacité de la régulation du marché de l'art en limitant les conflits d'intérêts, nous sommes convaincus que cette proposition de loi vont dans le bon sens nous mesurons aussi les limites de son action, nous devons poursuivre nos efforts pour relancer le secteur qui accuse un très fort déclin depuis 50 ans jusque dans les années 60 la France était au coeur du marché de l'art mondial aujourd'hui, les rapports de force économique et normatif ont changé et l'attractivité de la place de Paris arrive loin derrière, New-York, Londres et Hong-Kong cette partition récentes témoignent de la forte de compétitivité qui souffle sur le marché des ventes aux enchères désormais mondialisée volatile et fortement polarisé par des acteurs puissants tels que les maisons de vente Christie's et sothebys comment texte. Cliquez untel décrochage alors même que la France bénéficie d'un d'événements à dimension internationale, telle que la FIAC et d'un réseau de spécialistes de grande qualité, les objectifs de préservation du Patrimoine ont longtemps éclipsé les politiques de soutien au marché de l'art, la réforme du marché des ventes aux enchères engagées sous l'impulsion de la Commission européenne à partir des années 1980 a mis fin au blocage des commissaires-priseurs, opposé à toute forme d'évolution, les nombreux rapports publiés ces dernières années, témoigne à la fois de l'importance du secteur des ventes aux enchères et des difficultés rencontrées par le législateur pour le faire évoluer la loi du 10 juillet 2000 a opéré une première réforme libéralisant le marché français en mettant fin au monopole des commissaires-priseurs pour les ventes volontaires créant en même temps, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à l'origine, l'instance était essentiellement chargé de le délivrer des agréments aux opérateurs et de sanctionner les manquements à leurs obligations, explique libéralisation des ventes volontaires aux enchères publiques s'est poursuivie avec la réforme de 2011 autorisant notamment les commissaires-priseurs a effectué des ventes de gré à gré, malgré ces réformes, l'organisation du marché est restée archaïque et les divergences législative et réglementaire opèrent des distorsions de concurrence entre les différentes places de Paris, Paris, est en concurrence directe avec Londres au marché plus libéral et donc plus attractifs pour les Oeuvres, or il est difficile de se départir de règles qui limite tant bien que mal, fraude et opérations de blanchiment, il est aussi difficile à ce stade, de prévoir les conséquences certaines qu'aura le Brexit sur l'attractivité déjà faible de la place de Paris vis-à-vis de Londres sur le marché des enchères aussi le groupe les indépendants républiques et territoires apporte tout son soutien à cette réforme, nous invitons le gouvernement à poursuivre les efforts pour. Permettre à la place de Paris, non pas de retrouver son rayonnement d'antan car cela serait illusoire mais de s'affirmer face au Leadership du Royaume-Uni, nous avons un maillage de galeries exceptionnel des experts de très bon niveau, un savoir-faire reconnu et un réseau d'artistes contemporains qui ne demandent qu'à être Revel qu'être valorisé je vous Robert.

Monsieur le président, madame la ministre, hein. Madame la rapporteure à mes chers collègues, Paris, était autrefois la première place au monde pour les ventes aux enchères jusqu'aux années 70 la France est aujourd'hui en 4ème position, avec 5,6 pourcent de parts de marché, les États-Unis en détiennent 43 pourcent le Royaume-Uni 20 100 la Chine 19 pourcent. En croissance exponentielle sur la scène internationale, ce marché nécessite certes une surveillance mais aussi une fluidité accrue, ce constat n'est pas nouveau et, déjà, la loi du 20 juillet 2011 lois d'ailleurs adopté à l'initiative du Sénat avait assoupli la réglementation applicable depuis l'explosion de l'art numérique des nouvelles technologies de la demande asiatique a accru les exigences de rapidité et d'adaptation à ce marché très spécifique de biens meubles, les professionnels sont unanimes : le Conseil des ventes volontaires est aujourd'hui une structure trop lourde et trop rigide. La réforme portée ici par Madame Catherine Morin-Desailly, auteur de la proposition de loi et Madame Jackie de remédie rapporteur va dans ce sens, clarté simplification et professionnalisation tout en préservant une vraie régulation du marché. Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques devient ainsi le Conseil des maisons de vente sa composition assure une meilleure représentation des professionnels jusque-là le conseil était composé de 11 membres nommés par le gouvernement et qui pour la majorité d'entre eux n'appartenait pas à la profession, à savoir un membre du Conseil d'État de conseillers de la Cour de cassation, un membre de la Cour des comptes, 3 professionnels en exercice ou retraités, 3 personnalités qualifiées, un expert. Demain, le collège comprendra six, professionnels, élus par leurs pairs, un représentant du ministère de la justice, un représentant du ministère de la culture et 3 personnalités qualifiées nommées par la garde des Sceaux, ministre de la Justice a après avis des ministres chargés de la culture et du commerce, ainsi les représentants de la profession deviendrait majoritaire au sein du collège la fonction disciplinaire du Conseil appartiendrait désormais à une commission des différences et des sanctions indépendante du collège, le fait d'instituer un organe disciplinaire indépendant permettra à ce conseil d'être doté des moyens adéquats pour lutter contre le blanchiment de capitaux et les traffics illicites. Cette proposition de loi prévoit également que puissent être prononcées à l'égard d'un opérateur une sanction pécuniaire, alors que les sanctions disciplinaires applicables jusqu'à aujourd'hui était l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercer. Cela va dans le sens de sanctions plus efficace et individualisée. L'existence d'une autorité de régulation propres au secteur des ventes aux enchères est une spécificité française, réformer en profondeur cette autorité de régulation sans la supprimer apparaît aujourd'hui indispensable pour protéger efficacement vendeur et acquéreur et préserver l'image très positive dont bénéficient les maisons de ventes françaises à l'étranger, un système de régulation plus rigoureux constitue un Avantage certain au sein d'un marché mondial très compétitif, c'est pour cela que je vous invite mes chers collègues, tout comme notre groupe va le faire à soutenir cette proposition de loi, je vous remercie. Merci, la parole est maintenant à monsieur Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, et Madame la rapporteure et mes chers collègues, ce qui est intéressant finalement dans l'activité à laquelle nous nous livrons c'est que, à l'instar de certains grands écrivains que je ne citerai pas, mais que certains ici reconnaîtront nous cultivons le mode de la répétition, en effet, si l'on écoute les quatre discours ou 5 qui ont précédé et je suis sûr que de ne seront pas déçus par les 3 qui suivront, tout le monde dit qu'à peu près la même chose, ce qui est plutôt réconfortant mais ce qui fait que le ce qu'on appelle débat un côté. Tout à fait Herea rassurant finalement presque litanie vous voyez, a-t-elle écrivain je pense mes chers collègues, presque, dit Annick et donc je ne manquerai pas de dire, comme chacune et chacun de ceux qui m'ont précédé

J'ajouterai que le volume total des ventes aux enchères réalisée en France a progressé malgré quelques soubresauts, passant de 1 milliard 747 millions d'euros en 2003 à 3 milliards en 2018, mais cela n'a pas suffi à rattraper leur retard mondial alors Madame Morin-Desailly comme les autres orateurs, je veux lui rendre hommage, ainsi que Madame Jacky Deromedi car vous avez bien travaillé et le texte que nous étudions propose des modifications utiles, je dirais que celles-ci nous paraissent vraiment bienvenue, elle ne suffisent auront sans doute pas à rétablir des équilibres et à nous rendre une place que nous souhaiterions retrouver mais cela y contribuera Madame Morin-Desailly donc je tiens à saluer votre initiative, comme chacun l'a dit le Conseil des ventes volontaires deviendra le Conseil des maisons de vente et il aura pour mission de représenter la profession de l'accompagner dans l'exercice de son activité de vente Foch volontaires aux enchères de se positionner comme intermédiaires de confiance et comme relais d'information entre la profession, les pouvoirs publics et le grand public et d'organiser d'animer la formation des actuels et futurs professionnels des ventes volontaires. Il est heureux que l'on ait revu la composition du collège du Conseil des maisons de vente puisque le nombre de professionnels va être multiplié par 2, ce qui assurera un plus grande ancrage dans la profession. Et vous savez raison madame la ministre, il n'aurait pas été souhaitable que qui liait ès qualité des représentants du ministère de la justice ou du ministère de la culture, d'ailleurs, la commission des lois, l'a bien vu qu'il est revenu en arrière en disant qu'il y aurait des personnalités qualifiées, ce qui est tout à fait juste et ce qui évite une confusion des pouvoirs, qui eut été sachent bien, une fois que cela a été dit, je vais vous dire que je vais saluer le travail de la commission des lois, madame la rapporteure, puisque celui-ci, outre la modification dont je viens de parler sur les représentants des ministères auxquels auxquels on ne nous substituons Des personnalités qualifiées, il y a cette modification qui va maintenir l'obligation pour le Conseil des maisons de ventes de désigner un commissaire aux comptes et de secours soumettre au contrôle de la Cour des comptes, c'est une bonne mesure de même l'expulsion Express et Express de toute aide financière ou autre du Conseil des maisons de vente qui pourrait aboutir à du favoritisme. Enfin, le renforcement des prérogatives du conseil dans les domaines dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux du financement du terrorisme en lui confiant un pouvoir de contrôle sur place très bien notre groupe voudrait apporter sa contribution, cette contribution sera manifestée par 2 amendements qui sont d'ailleurs inspirés puisque comme mes prédécesseurs, je suis aussi très le rapport désormais célèbre de Madame Henriette chaud bon et de Me Édouard de Lamaze, qui va recevoir ici, monsieur le président de la commission des lois, une publicité inespérée donc cet excellent rapport. Il vise que les mais son de vente voies élargit leurs compétences soient leurs compétences élargies au inventaire successoraux facultatif, c'est-à-dire où s'inventèrent fiscaux, hé bien, nous vous proposons, mes chers collègues de retenir cette proposition. Nous avons fait d'eau, un autre amendement relatif à la terminologie parce que eux ils nous est appareil paru qu'il était mieux de désigner les choses telles qu'elles sont en parlant finalement de commissaires-priseurs puisque vous voyez que le terme de commissaires-priseurs judiciaire est appelée à disparaître à l'horizon 2023, donc parlons des commissaires priseurs et parlons des maisons de vente mais moi j'ai trouvé que c'était mieux d'appeler les choses par leur nom, plutôt que de maître par opérateur, vous savez, opérateur ça fait partie de ces mots-valises que l'on trouve partout, mais comme cela n'a pas eu l'air de vous plaire, madame la rapporteure, nous avons changé notre amendement pour marquer personne ça se discute, enfin, c'est un pas dans votre direction, toujours est-il que je conclurai comme je l'ai fait ce matin en commission en rappelant cette phrase d'Albert Camus : Mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde, je vous remercie de votre attention et nous voterons ce texte bien entendu. Merci monsieur Sueur. Hein madame la ministre, mes chers collègues, il est minuit passé de quelques minutes, je vous propose de prolonger notre séance afin de poursuivre et d'achever l'examen de ce texte, s'il n'y a pas d'observation. Il en est ainsi décidé donc la parole est maintenant à Madame Françoise Laborde. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il est rare que les parlementaires s'empare de la question du marché de l'art de sa régulation et incidemment de son avenir, il est vrai que pour les nombreuses esthète siégeant parmi nous, la notion même de marché de l'art est tabou pour les détracteurs d'une telle vision les Oeuvres ne sont pas des biens de consommation comme les autres, à l'instar de la conception de comptes pour qui le beau et l'objet d'une satisfaction désintéressée et libre, pour autant il existe évidemment un vaste marché des objets d'art dans les foires, les galeries, les salles de vente mais aussi désormais sur internet, l'acquisition d'Oeuvres d'art donne lieu à la rencontre du offre et d'une demande et à la formation d'un prix ce marché d'ailleurs considérables, comme le soulignait Stéphane Travert dans un intéressant rapport d'information publiée en 2016 l'apport dans le PIB français du secteur économique de la culture englobant le marché de l'art est devenu très important, il estimait ainsi que le secteur des arts visuels représenter à lui seul 21,4 milliards d'euros et 313000 emplois du côté des artistes cette réalité d'ailleurs produit des réactions ambivalentes, on pense à la provocation de Bansky ayant programmé la destruction d'une de ses Oeuvres en pleine vente ou à l'inverse, comme le fait Jeff Koons à la présentation assumer de comme un objet commercial peut-être le plus plus que sur les autres marchés, du fait de comportement d'ostentation de l'importante subjectivité de la perception du beau ou encore du rapport de l'artiste à ses mécènes, la formation des prix sur le marché de l'art reste un phénomène mystérieux, on s'étonne autant d'apprendre que certains artistes exposés dans nos musées nationaux ont connu des existences misérables que de constater la cote élevée d'artistes du mouvement global kitsch ou encore de la tendance des objets merveilleux, très en vogue chez les millionnaires de la planète, ce phénomène complexe de formation du prix est encore plus frappant dans l'art contemporain, comme l'écrivait l'historienne et sociologue de la Raymonde Moulin disparu cet été, l'art contemporain dépendait essentiellement du marché parce qu'il n'était pas compris ni acheté par les institutions, le marché français a longtemps fait la pluie et le beau temps des valorisations artistique internationale, s'appuyant sur des maisons de vente réputé sur des salons d'avant-garde et un important issues de mécènes et de galeries, mais l'âge d'or de la place de Paris est derrière nous, avec le recul des transactions opérées sur le sol français, ainsi, la France est progressivement passé de premières, places de vente à 4ème place à partir des années 60 pour 5 pourcent des parts du marché aujourd'hui, derrière les États-Unis, l'a déjà été dit le Royaume-Uni et la Chine, qui représente 83 pourcent du marché l'archaïsme des institutions historique du marché de l'art français est une des causes de ce recul parmi d'autres, la modernisation du statut de commissaire priseur est intervenu très tardivement, en 2000 puis en 2004, après la création du Conseil des ventes volontaires et l'amorce d'une régulation de ce segment du marché de la notre première réaction, et donc de regretter que cette proposition de loi ne recouvre pas un Champ plus vaste pour offrir des solutions plus variés à l'appui de son objectif, nous entendons qu'il existait depuis la loi Macron de 2015 des points à régler afin de permettre à la nouvelle profession de commissaires de justice de conseillers solide et sa mise en orbite d'ici 2022 en favorisant les meilleures conditions de rapprochement entre commissaire judiciaire et huissiers de justice, sans oublier les notaires qui est fluctue ponctuellement des ventes volontaires, nous avons d'ailleurs quelques propositions s'agissant de la nouvelle composition du conseil des maisons de vente et de la commission des sanctions afin d'en moins renforcer l'indépendance et l'intégrité nous aurons Luc, l'occasion de l'expliquer dans le détail, mais il nous paraît ainsi impertinent que la composition de ce conseil, prennent en compte des acteurs qui, sans être partie prenante au Ventoux volontaires puissent apporter leur expertise propre du monde de l'art en tant que représentant d'écoles ou de galeristes de la même manière, en août, prenant acte des constats du rapport travers nous souhaiterions que les professionnels des ventes volontaires représentant leurs collègues au sein du conseil ne soient pas tous issus du petit monde parisien, enfin, il s'agit d'une vigilance constante du groupe RDSE, à la suite des travaux de Jacques Mézard, nous sommes très attachés à ce que l'activité de régulation exercée par la commission des sanctions ne soit pas réservé aux anciens membres des plus hautes juridictions françaises mais puisse être ouverte à des profils plus divers recrutés sur base du mérite dans toutes les juridictions du territoire je redis en fait notre déception que ce texte ne puisse pas servir de véhicule législatif pour discuter d'autres sujets effectivement susceptibles de restaurer la place de l'influence artistique dans le monde, nous savons que nos concurrents disposent de leviers d'influence plus important pour soutenir les travaux de leurs artistes auprès des acquéreurs du monde entier, dont l'origine, c'est qu'on cible considérablement diversifié notre groupe considère pour sa part que la simple adaptation du régime des ventes aux enchères publiques ne suffira pas à rattraper le retard accumulé la spécialisation de nos maisons de ventes sur des segments de marché moins porteur que l'art contemporain, tels que le mobilier, ainsi que leur faible proactivité Allen ternational en sont aussi une cause majeure, sans doute faudrait-il réfléchir aux moyens de développer un meilleur soutien de nos institutions artistes contemporains français mais ce n'est pas le coeur de notre sujet en cette heure tardive, le groupe RDSE dans tous les cas ne s'opposera pas au bord au modernisation que ce texte entend réaliser, je vous remercie. Merci, la parole est maintenant à monsieur François Bonhomme pour 4 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le secteur des enchères est aujourd'hui fortement encadrés. Et la présence d'une autorité de régulation est à ce titre une singularité française, bien sûr, cette singularité ne manque pas d'être questionné la proposition de loi de notre collègue Catherine Morin-Desailly s'inscrit dans la continuité de la mission mise en place par Madame le garde des Sceaux sur l'avenir de la profession d'opérateurs de vente volontaires 41 propositions avaient été alors formulé pour encourager le développement d'un état d'esprit plus entreprenarial mais aussi ouvrir davantage activité des vannes volontaires cette proposition. inscrit dans cet objectif de réformer en profondeur le système français de régulation des ventes volontaires de meubles aux enchères en modifiant notamment la dénomination la composition, l'émission et le fonctionnement du Conseil des ventes volontaires naturellement j'y souscris pleinement et salue particulièrement les apports de la commission des lois pour préciser et compléter les dispositions proposées afin de poursuivre l'effort de mise à jour de notre législation et d'accompagner la transformation des maisons de ventes françaises dans un contexte de concurrence internationale de plus en plus féroce, je pense notamment à l'article 2 qui prévoit de rendre aux personnes qui tiennent marteau, le titre de commissaire priseur à compter du 1er juillet 2022, date de la création de la profession, commissaires de justice par regroupement des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires je pense aussi à l'extension du régime légal des ventes de meubles aux enchères aux mêmes incorporels les différentes mesures contribueront à réformer le système français de régulation des ventes aux enchères en ce sens, c'est une amélioration que nous saluons et que nous voyons favorablement. Mais cette amélioration ne doit pas nous empêcher de le resituer dans un contexte de bouleversement total du marché de l'art qui a abouti, ça l'a été dit au contournement du marché français. Les rapports annuels sur le marché de l'art mondial nous confirme année après année, les records d'adjudication quand on sait qu'il s'est construit plus de musée entre 2000 et 2019 que durant tout le XIXe et XXe siècles réunis, on comprend que seule industrie muséale, qui en est le moteur qui le moteur de ce marché et qui explique largement sa croissance spectaculaire et sans bouleversement, un marché où les artistes chinois qui représentent plus du quart de ce marché au détriment des artistes européens et français, un marché où toutes les maisons de ventes dans le monde sont aujourd'hui présentes sur Internet, alors qu'elle n'était songez songez-y que 3 pourcent en 2005, c'est une réalité que l'on ne peut ignorer cela fait certes bien longtemps que la France a dégringolé dans le classement mondial des 22 un cher quand la France détenait 50 pourcent du marché de l'art dans les années 50 contre autour de 5 pourcent aujourd'hui, sans parler de son rang anecdotique sur le marché de l'art contemporain, ce sont désormais les maisons chinoises, américaines et anglaises qui domine le marché Draw est un état de léthargie et observe impuissante Sotheby's et Christie's se développer tout cela permet de resituer la place réduite et malheureusement modestes de la France et de s'interroger aussi parfois sur le rôle quelque peu ornemental de l'État, en tout cas du ministère de la culture, on ne peut s'empêcher de penser à l'appréciation que porte l'historien d'art et conservateur du Patrimoine Jean clair sur la situation de l'art en France, il y a 20 ans. Jamais, disait-il, l'art n'aura joué de pareilles considérations officialité institution Maison de la culture musée: livres, revues biennale rétrospective Exposition géante foire vente aux enchères alimente son souvenir entretiennent sans regret exalte ses sursaut enregistré ces traces les plus minces de son agonie, il a ajouté : peu d'époque comme la nôtre, auront connu pareil divorce entre la pauvreté des Oeuvres qu'elle produit et l'inflation des commentaires que la moindre panne très de suscite, je ne suis pas sûr que cette situation est véritablement changé, en tout cas, elle nous permet de resituer les défis de la France, patrie de l'art, que la France doit relever concernant tant la place des artistes que la place des professionnels français sur le marché de l'art mondial, je vous remercie.

Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le Sénat examine aujourd'hui la proposition de loi déposée par le président, Catherine Morin-Desailly, cette proposition de loi refond le Conseil des ventes mot volontaires de meubles aux enchères publiques, dont la composition et les missions sont aujourd'hui inadaptés à la réalité du marché de l'art de l'avis de tous, cette réforme est indispensable pour que la place française retrouve une dynamique qu'elle a perdu au fil du temps, au point de faire de la France un acteur minoritaire s'du marché de l'art mondial pour ma part j'insisterai tout particulièrement sur la nécessité de veiller au bon fonctionnement de ce marché fortement exposée au risque de blanchiment ou de trafic illicite pour lutter contre ces dérives, le Conseil des ventes volontaires n'a jusqu'à présent joué aucun rôle, et pour cause, il ne dispose pas de compétences en matière de détection des dysfonctionnements du marché de l'art et c'est à Tracfin et à l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels qu'il revient de mettre à jour les dérives potentielles en matière de négoce, il est devenu d'autant plus urgent de se doter d'instruments de régulation que la place de Paris a été secouée, vous vous en souvenez certainement par des affaires retentissantes, qui n'a pas gardé en mémoire la triste affaire Aristophil dans laquelle pas moins de 18000 personnes petits épargnants ou investisseurs fortunés ont perdu près de 800 millions d'euros, les investisseurs étaient invités à acquérir des produits d'épargne constituée de part indivise de pièces autographes, lettres et manuscrits, avec la promesse d'un rendement annuel de l'ordre de 8 ce rendement était indexé sur la hausse du marché de ses biens en France, elles-mêmes artificiellement alimenté par l'intense activité d'achat de la société Aristophil, la bulle spéculative, comme cela était prévisible, a éclaté, des actions judiciaires ont été engagées et l'entreprise a été liquidé, le 4 août 2015, laissant derrière elle des investisseurs floués et le monde culturel en plein émoi, le marché de l'art, a été malgré lui, pris dans une tourmente qui a sérieusement entaché sa réputation, la dispersion de près de 130000 pièces est en cours, leur mise sur le marché nécessite de conjuguer 2 impératifs contradictoires, à savoir réaliser les collections dans des délais suffisamment courts pour que les épargnants puissent récupérer une part de leur investissement mais aussi suffisamment long pour éviter à ce marché étroit du manuscrit de s'effondrer, pardon, excusez-moi ont hélas fait ressortir une perte de valeur importante, ses ventes sont toutefois l'occasion pour les institutions culturelles de faire entrer dans leur collection des pièces importantes pour le Patrimoine national que parfois Aristophil les avaient empêchés d'acquérir à des prix raisonnables, certaines de ces pièces révèlent de la catégorie des archives publiques, il n'a, il y a, il n'est lié inaliénable et imprescriptible d'autres présentent un intérêt patrimonial exceptionnel et justifie une interdiction de sortie du territoire pas classement comme trésor national, c'est le cas de manuscrits, d'André Breton et du marquis de Sade retiré des ventes en 2017 quelques pièces possédant un intérêt patrimonial avéré mais non exceptionnelle ont rejoint des collections de plusieurs institutions culturelles, enfin une part importante des biens constituant les collections Aristophil ne présentent pas de réel intérêt patrimonial et une entrée dans les collections nationales n'est pas pertinente, 2 questions majeures d'or de public et doivent, de mon point de vue, être rapidement pour éviter que ne-t-elle à faire, se reproduise une question de surveillance des produits d'épargne, en effet, le contrat de placement était rédigé de telle manière que l'Autorité des marchés financiers, s'était déclarée incompétente à son corps défendant, et c'est la DGCCRF, qui avait dû instruire au titre de la tromperie au consommateur, une question de surveillance prudentielle du marché de l'art, et plus spécialement de la profession d'expert et sur ce dernier point, même si nous devons nous réjouir de la qualité du dispositif français encadrant l'expertise des progrès peuvent encore être réalisés concernant le titre d'expert notamment insuffisamment protégé l'accès à la profession le statut général encadrant son exercice la responsabilité et la nature des obligations des experts devront faire l'objet d'une réflexion approfondie à court terme, la nouvelle structure créée par la proposition de loi ici présente, pourrait en être le cadre, il en va de la stabilité de la qualité du marché de l'art, à l'heure où celui-ci draine des sommes d'argent considérables et attire de plus en plus d'investisseurs, je vous remercie. Merci, chers collègues, la discussion générale est Close, nous passons donc à la discussion du texte de la commission avant l'article 1er, nous avons une proposition d'articles additionnels : c'est l'amendement ne fructifier présenté par monsieur Jean-Pierre Sueur. Le le président, j'ai présenté cet amendement lors de mon intervention dans le débat chez General d'une part, sous la forme qu'il avait ce matin lors de sa présentation commission et sous la forme rectifié, que j'ai que je présente, pour des raisons que j'ai exposées. Merci madame la rapporteure, l'avis de la commission. Madame Madame le Ministre. Sagesse. Sagesse donc pas d'explication de vote donc je mets cet amendement on voit avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du gouvernement qui est. Pour. Qui est contre l'abstention donc. L'amendement est adopté, nous passons à l'article, l'article 1 avec l'amendement 10 rectifié, monsieur Jean-Pierre Sueur également. c'est un amendement de conséquence, Monsieur le Président. pour, avec 2 avis un favorable de sagesse qui est contre, abstention donc l'amendement est adopté, j'ai ensuite en discussion commune 2 amendements et un sous-amendement alors l'amendement numéro 2 du gouvernement, Madame la Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames siens triste, messieurs les sénateurs, l'amendement que je vous propose, précise que parmi les professionnels élus 3 devront exercer en Île-de-France et 3, hors Île-de-France, il vise à traduire ainsi : je l'ai expliqué dans mon discours tout tout à l'heure, il vise à traduire la diversité territoriale des opérateurs de vente volontaires parmi les opérateurs qui seront élus au sein du Conseil des maisons de ventes en 2017 59 pourcent des adjudications sont concentrées en Île-de-France et la forte concentration concentration des ventes représentent aussi finalement une fragilité pour le marché français, qui est exposé aux stratégies des sociétés multinationales et donc je pense que le maillage territorial des sociétés de vente volontaire, c'est une richesse le préciser également, il est important que la composition de l'instance de régulation reflète cette richesse territoriale. Merci madame la rapporteure le sous-amendement de la commission. La commission des Lois avait choisi comme le prévoyait la proposition de loi initial de laisser au pouvoir réglementaire, le soin de définir les modalités d'élection des représentants de la profession au sein du Conseil des maisons de ventes de manière à assurer la représentation de la diversité des opérateurs en terme de taille de structures et d'implantation géographique, le gouvernement nous propose en lieu et place de ce renvoi au décret d'inscrire dans la loi que les professionnels, élu au conseil devront exercer pour la moitié d'entre eux en Île-de-France et pour l'autre moitié sur le reste du territoire français, je constate que, d'après les statistiques rendues publiques par le Conseil des maisons de vente environ un tiers des opérateurs de ventes volontaires sont établis en Île-de-France l'Île-de-France concentre 61 pourcent du montant total des adjudications cette part étant en augmentation dès lors la répartition par moitié proposée par le gouvernement me paraît équitable, je m'interroge cependant sur l'opportunité de fixer cette répartition dans la loi ce qui est un facteur de rigidité, il faudra légiférer à nouveau si l'évolution du marché impose un jour de modifier cet équilibre malgré ces réserves, avis favorable sous réserve de l'adapter, de l'adoption du sous-amendement. Merci dans la discussion commune l'amendement numéro 6 rectifié Madame Françoise Laborde. Merci monsieur le président, madame la garde des sceaux, madame la rapporteure, mes chers collègues, cet amendement visait dans le même esprit que l'amendement de déposés par le gouvernement à diversifier la provenance géographique des représentants d'opérateurs des ventes volontaires au sein du Conseil nounours à Lyon, à la rédaction du gouvernement en attirant donc toujours l'attention sur la diversité géographique et notre intention étant satisfaite je retire mon amendement.

l'édition, je vous amendements. La vie sur sous-amendement et favorable. L'avis est favorable, très bien, donc je mets aux voix le sous-amendement de la commission avec un favorable du gouvernement qui est pour. pour. Et contres. Donc il est adopté, et maintenant je mets aux voix l'amendement du Gouvernement ainsi sous-amendé avec un avis favorable cette fois-ci de la Commission, donc qui est. Pour contre abstention. Donc que cet amendement est ainsi adopté l'amendement numéro 5 rectifié Madame Françoise Laborde. Merci monsieur le président, madame la garde des sceaux, madame la rapporteure, mes chers collègues, la présente proposition de loi modifie considérablement la composition du Conseil afin d'y renforcer la présence des professionnels du secteur, dont le nombre passe à 6 au lieu de 3 nous sommes vigilants à ce que ce conseil ne deviennent pas pour autant une instance ordinale et c'est pourquoi nous serions favorables à ce que certains postes de membres soit explicitement réservé à d'autres professions, compte tenu des constats dressés en 2016 par le député Stéphane Travert notamment l'intérêt trop tardive des maisons de vente pour l'art contemporain, aujourd'hui dominant sur le match, marché international, nous avons réfléchi à des moyens de sensibiliser les opérateurs de vente volontaire au courant artistique émergents permettre aux représentants des Eaux-Vives et de rencontrer un représentant des écoles d'art français et des galeries pour être un moyen indirect de satisfaire ce 2ème objectif, c'est pourquoi nous vous proposons cet amendement dont l'objet est, vous l'aurez compris de réserver un poste de membre du Conseil, un représentant des écoles supérieures d'art français et un représentant des galeristes, je vous remercie. Merci Madame Jackie Drôme dit d'avis de la commission. Cet amendement a pour objet d'élargir la composition du collège du Conseil des maisons de vente à un représentant de l'association nationale des écoles supérieures d'art, un représentant des galeries d'art, je n'y suis pas favorable pour pour plusieurs raisons : tout d'abord le conseil des maisons de vente est une autorité de régulation d'une activité professionnelle, il n'y a pas de raison d'y faire siéger ès qualité des représentants du monde académique ou d'une autre profession celle des galeristes bien sûr des échanges doivent avoir lieu entre ces différents secteurs, mais l'enceinte appropriée pour ces échanges n'est pas une autorité de régulation ensuite l'amendement aboutirait à déséquilibrer la composition du collège du Conseil des maisons de vente puisque les représentants de la profession, il redeviendrait minoritaire, enfin, l'association nationale des écoles supérieures d'art n'a aujourd'hui aucun fondement légal ou réglementaire et il ne me paraît pas opportun de consacrer son existence dans la loi : avis défavorable. Merci madame la ministre avait du gouvernement. Monsieur le président, madame la sénatrice, je partage l'avis de Madame la rapporteure, j'ajoute que l'on pourrait imaginer, sinon souhaiter une compétence cette nature-là l'inclure dans les personnalités qualifiées qui pourraient siéger je ne pense pas qu'il soit pertinent de la désigner es-qualité avis défavorable. Merci à l'amendement est retiré. Oui, je retire, puisque j'ai une réponse sur les experts et sur la régulation, je je retire cet amendement. Merci donc l'amendement est retiré l'amendement suivant : c'est l'amendement numéro un du gouvernement amenuise. amenuise. Le président, mesdames, dessinatrice, messieurs les sénateurs, c'est un amendement qui vise à modifier le mode de désignation du président du Conseil des maisons de vente, l'amendement prévoit que ce dernier est nommé par le garde des Sceaux, ministre de la justice, parmi les personnalités qualifiées et non parmi l'ensemble des membres du nouveau Conseil des maisons de vente, comme le prévoit la proposition de loi j'ai expliqué les raisons pour lesquelles je vous proposer cette modification dans mon propos introductif, il me semble que si la présence accrue des professionnels au sein du Conseil des maisons de vente répond à une demande légitime et ancienne des professionnels, il est toutefois nécessaire de préserver un équilibre entre le caractère professionnel du Conseil et sa fonction de régulation et il ne m'apparaît en effet nécessaire d'éviter que la présence majoritaire des professionnels au sein du Conseil des maisons de vente rapproche cette autorité d'un ordre professionnel, alors que nous voulons faire une autorité de régulation et donc il me semble, à ce titre que le choix du président du Conseil parmi les personnalités qualifiées et plus judicieux et mieux adaptée à ce que nous voulons faire de cette instance. Merci madame la rapporteure, la ville des commissions. Cet amendement prévoit que le président du Conseil des maisons, des maisons de vente soit choisi parmi les non-professionnels qui siègent au sein du collège, le gouvernement fait valoir que le rééquilibrage de la composition du collège où les professionnels deviendraient majoritaires justifie, eu égard à la mission de régulation du Conseil que son président soit je cette parmi les non-professionnels, c'était l'argument que nous pouvons entendre, néanmoins, il serait également souhaitable que le président du Conseil des maisons de vente et lui-même l'expérience des ventes aux enchères, cela ne peut que faciliter l'exercice de sa mission, madame la garde des Sceaux, je vous propose une solution de compromis, la proposition de loi dans sa rédaction actuelle prévoit que le président du Conseil soit nommé sur proposition du collège, pourquoi ne pensent ne pas se contenter de supprimer ce pouvoir de proposition, dès lors, vous et vos successeurs seriez entièrement libre de choisir le président parmi parmi les membres du collège, qu'il s'agisse des représentants élus de la profession ou des personnalités qualifiées nommées par arrêté ministériel, la commission donnerait un avis favorable à cette rédaction, à défaut, nous préférons que le débat se poursuive au cours de la navette.

Madame le Ministre. Je vous remercie madame la rapporteure de la manière dont vous avez présenté, à la fois l'intérêt de mon propre amendement mais également la solution de modifications que vous proposez comme je l'ai expliqué tout à l'heure je je comprends très bien l'évolution que vous faites, puisque vous enlevez le fait que la nomination par le garde des Sceaux, enfin vous vous souhaiteriez me proposer que la nomination par le garde des Sceaux se fasse indépendamment de toute proposition du collège, donc je considère effectivement que c'est un un, un point important, mais toutefois vous maintenez l'intérêt que le président puisse avoir une expérience notamment des ventes volontaires, je vous le redis et en comprenant parfaitement votre position, je ne pense pas que cette solution-là soit la meilleure, elle ne me semble pas la meilleure, puisque moi je considère que le président doit pouvoir être à distance finalement de ce qui est le quotidien de, de, de, de ces praticiens et que il ne faut pas aller vers ce qui pourrait entraîner une confusion avec un ordre professionnel pour cette raison, je préfère m'en tenir à l'écriture, que je vous proposais et donc je ne souhaite pas aller dans le sens où la modification que vous suggérez. Merci donc c'est un avis défavorable de la commission, monsieur Jean-Pierre Sueur, explications de bottes. monsieur le Président notre groupe sera contre cet amendement, madame le Garde des Sceaux, en dépit des efforts accomplis par madame le rapporteur et que je salue, en effet, je trouve que votre vision est quelque peu passéiste par rapport à cette organisation, madame le Garde des Sceaux et venant de vous, cela m'étonne quelque peu je voulais signaler mais c'est évident que ce que vous proposez, peut se traduire par un blocage institutionnel, si le président du conseil de la maison de vente nommés par le garde des Sceaux n'est pas en phase avec les professionnels qui seront désormais majoritaire au sein du collège, il y aura bien sûr un problème et il nous apparaît que mieux vaut rester dans un souci démocratique à la rédaction actuelle, à savoir que le président du Conseil des maisons de vente est nommé par le quart de des Dessau sur proposition des membres du collège qui pourront voter pour, si en leur sein un repos un précédent. Merci Madame Catherine Morin-Desailly, explications de vote. Oui je je remercie mon collègue d'apporter quelques éclaircissements finalement la proposition que j'avais initialement formulée dans la la proposition de loi, je dois dire que je m'étais aussi inspiré de cet excellent rapport qui est le rapport de monsieur de la base et de madame Chaumont qui pointé du doigt le fait qu'en effet il y avait pas de raison à priori d'exclure quelques membres, que ce soit comme pouvant être potentiellement désigné comme président du du Conseil des ventes bien entendu madame la garde des Sceaux, la navette sera aussi l'occasion d'approfondir le dialogue, la réflexion sur ce sujet, mais en effet, nous voulons une comment dirais-je avancer vers la modernisation de la régulation, c'est bien le type de la proposition de loi et le mode de désignation aussi de l'autorité fait partie des réflexions engagées. Merci donc je vais mettre aux voix cet amendement du gouvernement avec un avis défavorable de la commune. Sion, qui est pour. Qui compte. Abstention donc il n'est pas adopté l'amendement suivant le 7 rectifié et Madame Françoise Laborde. Merci monsieur le président, madame la garde des choses madame la rapporteure, mes chers collègues, vous le savez, la question de la nomination des membres des instances de régulation est un sujet de préoccupation du groupe RDSE, comme je l'ai déjà dit depuis leur rapport d'information de Jacques Mézard consacré aux autorités administratives indépendantes, en effet, bien que l'on ait tendance à minimiser la portée de ces nominations, elles sont d'importance, d'abord parce qu'ils traduisent l'influence parfois démesurés de certains corps au sein de nos institutions, au point de se réserver telle ou telle position clé au sein de l'État, sans possibilité de contrôle pour les autorités politiques, ensuite parce que cette influence s'exerce au détriment d'autres corps qui seraient également compétent pour exercer ses fonctions en quelque sorte les fonctions réservée à certains corps amenuise les perspectives des autres et Alter donc le principe de carrière et de valorisation du mérite républicain tout au long de cette carrière enfin parce que la mainmise d'un corps sur ses fonctions de régulation renforce les risques de conflit d'intérêts, lorsque ce même corps se voit également ouvrir d'importantes perspectives professionnelles dans le secteur qui est appelé à réguler pour toutes ces raisons, déjà exprimé, nous sommes favorables à une révision des conditions de nomination au sein de la commission des sanctions nous souhaitons que celle-ci soit ouverte aux magistrats de l'ordre administratif et judiciaire exerçant dans les juridictions de 1er et second degré se pose également la question de l'autorité chargée de proposer les candidats à ces fonctions, alors que dans la rédaction, l'autorité de nomination est lié par cette proposition, la rédaction proposée n'est donc pas satisfaisante puisque dans les 2 ordres, elle confie ce pouvoir à une seule personne, lui conférant des pré-Gora des prérogatives démesurées, nous serions donc favorable à ce que cette émission revienne dans un cas au Conseil supérieur des Trabis tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, présidée par le vice-président du Conseil d'État et dans l'ordre judiciaire, à ce que cette proposition soit formulée par le Conseil supérieur de la magistrature ce par souci d'équité entre les membres de ces différents corps et par souci d'indépendance de la commission des sanctions, je vous remercie. Merci madame rapporteur l'avis de la commission. Cet amendement prévoit de modifier la composition de la commission des sanctions du Conseil des maisons de vente, l'amendement a pour objet d'un côté, d'élargir le vivier à l'ensemble des magistrats administrative ou judiciaire afin, je cite, de réduire la pratique des emplois réservés aux grands corps, d'un autre côté, de réduire le vivier en le limitant au musée au magistrat ayant exercé depuis plus de 10 ans et en supprimant la faculté de nommer des magistrats honoraires je comprends l'intention d'élargir les perspectives de carrière des magistrats administratifs ou judiciaires qui n'ont pas le bonheur de servir au Conseil d'État ou à la Cour de cassation je comprends moins celle d'exclure par principe les magistrats honoraires dans sa rédaction initiale, l'amendement posait en outre des difficultés juridiques, par souci de consensus, la commission des Lois avait donné un avis favorable à l'amendement, sous réserve qu'il soit rectifié pour ne retenir que l'élargissement du vivier des personnes proposa je constate que la rectification opérée ne répond pas à cette demande, c'est donc un avis défavorable. Merci madame la ministre, l'avis du gouvernement. personne qui pourrait être membre du Conseil des maisons de vente toutefois, je pense, comme vient de le souligner, Madame la sénatrice de qu'il y a une difficulté de nature constitutionnelle puisqu'au fond vous ajouter aux compétences du CSM notamment et donc ça ne peut pas se faire par un simple texte de loi mais qu'il faudrait une loi constitutionnelle ou bien une loi organique à tout le moins, donc je crois qu'il nous sommes là face, une vraie difficulté pour ces raisons, je sollicite le retrait de votre amendement, à défaut, j'émettrai un avis défavorable. Merci Madame Laborde vous maintenez l'amendement. mais j'avais envie quand même qu'on en débatte à ma façon, si je peux me permettre et c'est pour ça que je n'aimais qu'une modification parce que quelquefois les membres honoraires sont un peu aussi dans l'ancien temps, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, donc je voulais du recul donc 10 ans au moins, mais pas spécialement un membre honoraire qui n'exerce plus, c'est pour ça que j'ai voulu présenter cet amendement de a même façon mais je maintenant je le retire, puisque de toute façon il aura un vote négatif. Merci d'amendements suivants : l'amendement numéro 15 madame Jacques Hydro-Mehdi pour la Commission. C'est un amendement de précision par cohérence avec l'adoption des amendements numéro 9 et 10 de monsieur Sueur

Avis favorable, Monsieur le Président. Avis favorable donc je mets aux voix cet amendement de la commission avec un avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre, abstention, donc il est adopté, le 16 madame Deromedi coordination.

le 17 Madame Jacques Hydro-Mehdi. Cet amendement vise à compléter les dispositions transitoires en vue de la création du Conseil des maisons de vente.

Qui est contre l'abstention, donc il est adopté, je mets maintenant aux voix, l'article 1er qui est pour l'article 1er. Contre, abstention. Il est adopté article additionnel après l'article 1er amendement 11 rectifié bis monsieur Jean-Pierre Sueur. Merci monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il s'agit d'appliquer la recommandation numéro 5 de l'excellent rapport déjà cité de Madame Chow bon et de monsieur de la base qui propose donc dans cette recommandation. De permettre aux maisons de vente c'est élargir leurs compétences aux inventaires successoraux facultatif, c'est-à-dire où s'inventèrent fiscaux. Merci l'avis de la commission madame la rapporteure. Cet amendement a pour objet d'habiliter les opérateurs de vente volontaire a réalisé les inventaires dit fiscaux comme vous le savez la loi ou le règlement impose dans certains cas de réaliser l'inventaire d'une succession lorsque l'un des heures et des héritiers accepte la succession à aux à concurrence de l'actif Net lorsque la succession est vacante lorsque les scellés de succession sont levés, alors que toutes les parties ne sont pas présentes ou représentées et qu'elles n'ont pas donné leur accord pour une levée sans inventaire en dehors de ces hypothèses, la réalisation d'un inventaire successoral est facultatif, il est alors réalisée dans les conditions et dans les formes prévues par les articles 13 29 et les suivants du Code de procédure procédure civile à l'inventaire peut ainsi être réalisé pour échapper à l'évaluation forfaitaire des meubles me blanc prévue à l'article 764 du code général des impôts en commission monsieur Sueur a proposé de rendent les opérateurs de vente volontaire compétent pour réaliser l'ensemble des inventaires successoraux, je m'y étaient opposé en revanche pour ce qui est des inventaires facultatif, notamment lorsqu'ils sont établis à des fins fiscales il est envisageable qu'il puisse être réalisé par des opérateurs de vente volontaire, le ministère de l'Économie et des Finances, m'a fait savoir qu'il n'y était pas opposé le plus satisfaisant pour la cohérence du droit serait que le gouvernement étende par décret aux opérateurs de vente volontaire, la faculté de réaliser l'ensemble des et des inventaires successoraux facultatif en modifiant à cet effet, le code de procédure civile que l'article 764 du code général des impôts soit ensuite modifié pour envoyer aux formes prescrites par les inventaires obligatoire ou facultatif l'amendement de monsieur sueur se concentre sur la procédure applicable en matière fiscale, en attendant d'en savoir plus sur les intentions du gouvernement, je donne un avis de sagesse. Merci madame la ministre à l'avis du gouvernement. Merci monsieur le président, c'est effectivement un avis très favorable que je donne à l'amendement proposé par monsieur Jean-Pierre Sueur je crois que cet élargissement de compétences est tout à fait bienvenue et pour répondre à Madame la rapporteure de Khomeiny, il y aura effectivement des dispositions réglementaires qui devront devront être prises par la suite pour compléter la disposition législative que vous adopterez, je l'espère et tout ça est évidemment déjà prévu par la direction des affaires civiles et du Merci donc je vais mettre cet amendement on voit donc avec un avis madame la rapporteure Anne avis sagesse un avis de sagesse de la commission, un avis favorable du gouvernement. Qui est pour, qui est contre l'abstention. Donc, l'amendement est adopté l'article 2 amendements, numéro 3 du gouvernement ne le Ministre. Cet amendement Monsieur le Président, modifie la date d'entrée en vigueur de la modification du titre de commissaire priseur des ventes volontaires par celui de commissaire priseur des suggestions qui avait été fait précédemment dans le cadre de la réforme des commissaires de justice, les commissaires-priseurs judiciaires pourront utiliser leurs titres jusqu'au 1er juillet 2026 date de la suppression de la profession et donc afin d'éviter toute confusion entre le titre de commissaire priseur et du commissaires-priseurs judiciaire, il me semble préférable Duferco ainsi coïncider les 2, date d'entrée en vigueur au 1er juillet 2026. Merci madame la rapporteure, l'avis de la commission favorable donc, l'avis favorable de la commis. Si on donc je mets aux voix cet amendement du gouvernement avec un avis favorable de la commission qui pour. Compte. Abstention donc il est adopté, je mets aux voix, l'article 2 qui est pour l'article 2 contres abstention il est adopté, même vote pour l'article 3 même votre pour article 4 alors maintenant l'article 5 l'amendement 12 rectifié bis monsieur Jean-Pierre Serre. Ce le président c'est un amendement de conséquence, comme d'ailleurs l'amendement cathos rectifié bis. Madame Madame la rapporteure avis favorable Madame la Ministre, sagesse il. Favorable donc que je mets aux voix cet amendement avec 2 avis favorable qui est pour. Compte abstention donc. Il est adopté, vous m'avez indiqué que non, le 14 c'est pas le même, alors maintenant nous avons le l'amendement numéro 18 de la commission madame ne remédie. Coordination précision. Madame la Ministre favorable. Favorable, donc je le mets au. Voix qui est pour compte abstentions. Il est adopté, la demande l'amendement 13 rectifié, monsieur Jean-Pierre Sueur. amendement de conséquence favorable sagesse sagesse donc je mets aux voix, cet amendement avait qu'un avis favorable de la commission, un avis de sagesse du gouvernement qui est. Pour compte. Abstention est adopté.

Compte. Abstentions : l'article 5 est adopté l'article 6 amendements 14 fructifier bis amendement de conséquence Madame la rapporteure. Sagesse.

je mets aux voix, l'article 6 qui est pour l'article 6 contre, abstention est adopté, même votre article 7. Même vote pour l'article 8. Alors ensuite article additionnel après l'article 8. En discussion commune c'est un amendement et un sous-amendement l'amendement numéro 4 du gouvernement, Madame la Ministre. monsieur le président, c'est un amendement de transposition d'un texte européen, la Commission européenne a en effet adressé à la France le 20 juillet 2018, une mise en demeure, puis ensuite un avis motivé, le 7 mars 2019 pour mauvaise transposition de la directive 2005 36 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, si la dite directive qualification professionnelle, cet avis motivé et la dernière étape avant une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne parmi les griefs qui sont adressés à la France par la Commission européenne figure la non-transposition de l'accès partiel à la profession d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques l'accès partiel est issu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union, il permet à un professionnel pleinement qualifié d'exercer une partie seulement des actes qui relèvent d'une profession à part entière, en France, cette faculté, elle est encadrée dans des conditions extrêmement strictes et par un examen au cas par cas des demandes qui pourrait être refusée pour un impérieux motif d'intérêt général, cette transposition permettra donc au cas par cas et sous certaines conditions aux ressortissants des États membres de l'Union d'exercer en France, une partie de l'activité d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, par exemple la vente aux enchères automobile ou bien d'art asiatique, cet amendement vise ainsi à mettre notre législation en conformité avec la réglementation européenne et à éviter une saisine de la Cour de justice de l'Union. Merci donc j'ai un sous-amendement de la commission madame Jacky Deromedi. C'était l'avis favorable sous réserve de l'adoption de du sous-amendement.

Très bien, donc je mais s'il y a pas d'explication de vote je mets aux voix le sous-amendement avec un avis de sous-amendement de la commission avec un avis favorable du gouvernement qui est pour. Contre. Abstention : le sous-amendement est adopté, je mène maintenant aux voix l'amendement du Gouvernement ainsi sous- amendé avec un avis favorable de la commission qui est pour.

Oui Madame Catherine Morin-Desailly. En parce que l'heure est tardive, monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, juste pour remercier l'ensemble des sénateurs présents à cette heure tardive, qui ont contribué à enrichir le texte initial, c'est ensemble que l'on peut avancer vers des textes utiles et Madame Lagarde et sauce, c'est le but de cette proposition de loi, c'est en faire un texte utile qui va trouver aussi sa vie dans le cas de de la navette et j'espère qu'on arrivera à un accord qui nous permettra de répondre aux professionnels qui sont dans l'attente, comme je l'ai dit tout à l'heure, je voulais dire à ma chère collègue de la Commission de la culture, Françoise Laborde, que comme j'ai dit dans mon propos liminaire, l'objectif de cette proposition de loi n'était en aucun cas prétendent vouloir restaurer la place de la France et de sa compétitivité dans le marché là à l'international, je n'aurais pas cette prétention, je renvoie aux conclusions de la table ronde que nous avons tenu en mars 2018 avec la commission des Lois où là, nous avions évoqué un certain nombre de propositions propositions qui n'étaient pas or législatif mais plutôt réglementaire, fiscal, etc, la proposition de loi n'avait d'autre que Bute très modeste de moderniser la régulation du marché de l'art, je tiens à le dire pour répondre aux reproches qui m'ont été faits à la à la tribune, c'était pas l'objectif à atteinte, j'aurais pas eu cette prétention n'est-ce pas cher François Bonhomme voilà, merci en tout cas aux uns et aux autres bien sûr, je voterai ce texte ainsi précisé et enrichi. Merci madame Françoise Laborde, explications de vote. Oh ben oui parce que je vais le voter, nous le vote en touche et nous sommes là à une heure tardive, donc la modestie n'était peut-être pas ma qualité principale, ce soir, mais si on peut pas se régaler et port et pousser un peu le bouchon, c'est pas la peine qu'on soit là d'ailleurs, nous ne sommes pas oui. Merci, pas d'autres explications de vote. Donc je je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l'art qui est pour. Qui est contre, abstention. ce projet de cette proposition de loi est adopté. Mes chers collègues, je vais lever la séance, la prochaine séance, jeudi 24 octobre à 10 heures prendre pour l'examen de la proposition de résolution relative à la consolidation du pouvoir de dérogation aux normes attribué au préfet la séance est levée.